Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, je vérifie qu'il n'y a pas d'observation. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour. Pardonnez-moi, appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et interdire le démarchage de ses titulaires qui aura demande du groupe Rassemblement démocrates, progressistes et indépendants. Nous ouvrons la discussion générale avec la parole à la ministre. Carole Granjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.

Je souhaite en 1er lieu remercier le groupe RDPI et le CNR taire le sénateur Martin lévrier pour avoir inscrit à l'ordre du jour réservé à son groupe. Cette proposition de loi. Je tiens à saluer le travail effectué par Catherine Fabre qui s'était saisi avec détermination, de cette question pendant le quinquennat précédent. Il avait déposé une proposition de loi qui a constitué le socle sur lequel le texte a été bâti. Je suis donc très heureuse en tant que que Ministre de délégué chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle de soutenir aujourd'hui cette proposition de loi. La lutte contre les abus et la fraude au compte personnel de formation et un objectif qui doit tous nous réunir. C'est dans cette perspective que les députés de l'Assemblée nationale ont adopté ce texte à l'unanimité, avec le soutien du gouvernement. Je suis certaine qu'il recueillera à nouveau un très large consensus sur les bancs de cette assemblée. J'aimerais d'abord revenir sur le contexte d'examen de cette proposition de loi qui est une réponse ferme au détournement du compte personnel de formation. Le CPF fête cette année ses trois ans. Ce dispositif a rencontré un succès. Populaire incontestable auprès des Français. Près de 95% des actifs connaissent ça Tutti et environ 20% d'entre eux ont ouvert leurs droits depuis sa création en 2019. Il est autant mobilisés par les femmes que par les hommes. Il est davantage utilisé par les employés et les ouvriers que par les cadres incontestablement le CPF a véritablement faciliter la démocratisation de l'accès à la formation. Le CPF se retrouve à tous les carrefours de la vie professionnelle des Françaises et des Français, il est l'outil qu'ils peuvent mobiliser dans tous les moments charnières de leur vie pour préparer leur parcours professionnel se former à la création d'entreprise ou encore faire un bilan de compétence. Cependant. Ce succès massif du CPF a aussi ouvert la porte à des pratiques commerciales agressives voire abusives. Ces dérives consiste souvent à forcer les individus à acheter des formations contre leur gré ou de manière insuffisamment réfléchies. Cela s'est traduit par des appels des SMS ou des courriels intempestifs de la part de centres d'appel ou d'organismes de formation. Ces arnaques véhiculées bien souvent des informations erronées sur les droits de l'individu et sur l'objectif réel poursuivi par l'organisme. Les fautes graves telles que l'usurpation d'identité ou le détournement des droits du compte personnel de formation font l'objet d'un contrat contrôle accu accrue par la Caisse des dépôts et des consignations. Le préjudice financier lié aux pratiques abusives et frauduleuses est évalué à 43 millions d'euros en 2021, une somme qui a été multiplié par 5 en un an. Ce démarchage agressif nuit aux finances à la confiance et à l'image de l'outil et appelle une réponse ferme.-- Le gouvernement a agi pour mettre un terme à ces pratiques qui mettent en péril la lisibilité et la crédibilité du dispositif un renforcement du niveau de sécurité de la plateforme mon compte formation a d'abord été mis en place le 25 octobre dernier tout achat de formation est désormais sécurisé via le nouveau service France Connect plus ce service propose une authentification renforcée via l'application d'identification numérique de La Poste. Cette authentification renforcée permet de limiter les risques d'usurpation d'identité. Il s'agit bien d'un changement notable en terme d'usage pour les Français. Le réseau de la Poste et les maisons France services sont mobilisés pour accompagner les Français dans ses démarches. Avant même cette nouvelle phase de sécurisation techniques des actions de contrôle accru avaient déjà été menés pour améliorer la qualité de l'offre de formation. Le gouvernement a en effet envisager des mesures de régulation du secteur pour faire monter en qualité l'offre accessible par mon compte formation, je pense notamment à l'entrée en vigueur du Label Kaliopie depuis le 1er janvier visant à renforcer l'exigence de qualité, par les organismes de me de formation qui sont aujourd'hui près de 17.000 sur la plateforme contre 24.000 auparavant. Un travail particulièrement exigeant, a également été menée sur le renouvellement du répertoire spécifique qui a conduit à éliminer de tiers de certification dont l'intérêt n'était plus avéré pour l'évolution professionnelle des actifs. Enfin il y a quelques mois, sur demande de l'État c'est l'intégrité de l'intégralité de l'offre portant sur la création et la reprise d'entreprise qui a été revu par la Caisse des dépôts, près de 60% des offres ont ainsi été déréférencé car elles étaient apparus non conformes. Aujourd'hui plus personne ne peut dire que le compte personnel de formation rime avec formation de loisirs. Nous nous sommes donné les moyens de proposer un catalogue de formation utile pour l'emploi la professionnalisation et à monter en compétences, les actifs de notre pays. Il nous faut donc à présent oeuvrer pour éradiquer la fraude et le démarchage abusif de la plateforme. Cette proposition de loi vient donc renforcer plus encore l'arsenal de régulation. L'article 3 de cette loi prévoit une procédure de vérification des organismes de formation qui demande à être enregistrées par la plateforme. L'objectif est de garantir aux titulaires du compte que les organismes et la formation suivie remplissent bien tous les deux les critères d'éligibilité du compte personnel de formation, il permettra en août de garantir la qualité et l'honorabilité des organismes de formation inscrits sur la plateforme qui devront être à jour de leurs obligations sociales et fiscales. L'article IV de la proposition de loi introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale propose quant à lui une étape supplémentaire afin que les sous-traitants soient eux aussi soumis aux mêmes exigences que l'organisme de formation donneur d'ordres. Soyons clairs sur ce sujet. Il ne s'agit pas d'interdire la sous-traitance ni d'entraver la liberté de commerce mais nous constatons aujourd'hui que certains organismes de formation pourtant des référents pourtant référencé pardon sur la plateforme propose seulement ce qu'on appelle un portage Kaliopie. Je le dis clairement, ces organismes de formation agissent comme des sociétés écrans. Il s'agit. Ils savent que la Caisse des dépôts et des consignations ne peut ni identifiée, ni contrôlée. Les sous-traitants cet angle mort et donc un y a fraude potentielle, cette pratique n'est plus admissible et doit être régulée. Cette mesure a ainsi pour objectif d'assainir toute la chaîne de valeur en rendant les organismes de formation transparent et responsable vis-à-vis de leurs sous-traitants. L'article 4 1 prévoit un décret qui sera pris en concertation avec les représentants du secteur de la formation professionnelle pour préciser les modalités d'application de la disposition. Cette concertation a déjà démarré sous l'égide de mon cabinet depuis plusieurs semaines maintenant. Je tiens ici à rassurer les professionnels du secteur de la formation et en particulier les formateurs indépendants une attention toute particulière sera portée aux formateurs individuels qui sont des acteurs essentiels à la formation professionnelle. Nous ne pouvons pas décemment en effet leur demander les mêmes exigences que pour les organismes de formation qui occupe l'ensemble de la chaîne de la formation et qui dégage un chiffre d'affaires conséquent. Notre objectif est donc de protéger les citoyens qui souhaitent souscrire à une formation via via leur CPF en leur permettant de vérifier à qui ils ont à faire et en s'assurant de la qualité de l'organisme qui proposera la formation.-- Je veux dire ici toute la détermination du gouvernement à empêcher tout détournement du droit fondamental d'accès à la formation, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui nous donnera des leviers efficaces pour mieux prévenir lutter et sanctionner les abus et les fraudes au compte personnel de formation. Elle va en effet permettre d'interdire le démarchage abusif et de sanctionner plus efficacement. Ceux qui le pratiquent, y compris sur les réseaux sociaux en ligne. Nous ne pourrons que nous satisfaire de voir disparaître de tels abus. Plus d'influenceurs promettant monts et merveilles. Tablettes et smartphones plus de messages inacceptable incitant au recours au compte personnel de formation pour mieux le détourner de sa fonction initiale et l'instrumentaliser. Les amendes seront en effet très dissuasive jusqu'à 75.000 euros pour une personne physique et et 375.000 euros pour une personne morale. À la suite de publication illicite de la part de plusieurs influenceurs à propos des d'offres CPF. J'ajoute que la Caisse des dépôts et consignations a également saisi un cabinet d'avocats pour adresser des mises en demeure aux individus concernés. Un bon nombre d'entre eux, il y a déjà, d'ores et déjà répondu en s'engageant sur 3 points. L'arrêt de toute publicité en lien avec le CPF. La mise à disposition de documents des sociétés avec ils étaient en lien afin de de mener les enquêtes est effectué, le cas échéant, des dépôts de plainte et la publication sur leurs réseaux sociaux d'un message rectificatif. La proposition de loi va également dans son article de donner les moyens au de partager les informations dont il dispose pour mieux conduire la lutte contre la fraude. J'insiste sur cette nécessaire coordination entre les services de l'État et les opérateurs. Elle est absolument incontournable pour pouvoir resserrer les mailles du filet, vérifier les identités des suspects contrôler les habilitations à former traquer les fausses domiciliations et cetera. Nous devons en effet impérativement croiser les fichiers et les informations pour lutter efficacement contre les fraudeurs les traquer et les arrêter. C'est tout le sens de ce texte que je à qui je veux donner plus de moyens pour donner aux services de l'État, à la Caisse des consignation des dépôts et consignations ou encore à Tracfin, des moyens pour pouvoir identifier les fraudeurs et ne laisser aucun délit impunis. L'article 2 bis vise également à renforcer les pouvoirs de la Caisse des dépôts en lui accordant la capacité de recouvrer plus rapidement les sommes indument perçues ce pouvoir d'intervention directe et rapide sans saisine préalable de la juridiction administrative améliorera l'efficacité de la lutte contre l'évasion des fonds des fonds Mesdames, et messieurs les sénateurs, mais admise messieurs les sénatrices. Vous l'aurez compris, je crois que nous pouvons nous satisfaire du travail. Collectivement, réalisée sur ce sujet et transpartisan et véritablement d'intérêt général. Notre responsabilité est de protéger le CPF pour bien, pour le bien de nos concitoyens. Car protéger le CPF c'est protéger finalement la capacité des Français à se former ses protégés une application qui fait désormais partie de leur vie quotidienne, c'est protéger un droit qui se sont appropriés massivement grâce à la désintermédiation permise par cette application. Le CPF rappelons-le a rendu plus réel et plus tangible, la liberté de chacune et chacun de choisir son avenir professionnel et de maîtriser son parcours de vie en interdisant le démarchage abusif et en luttant mieux contre les fraudes nous redonnons toutes ses marges de manoeuvre au CPF et nous permettront à tous les actifs d'être en capacité de réussir cette transition professionnelle. Nous devrons prochainement compléter cette action de régulation du CPF en faisant en sorte qu'il soit mieux ciblées vers les besoins réels de l'économie, c'est-à-dire vers les métiers en tension ou les métiers d'avenir. C'est une réflexion que je vais mener en concertation avec les partenaires sociaux que je reçois aujourd'hui pour qu'il nous présente avec Olivier Dussopt la synthèse de leurs travaux paritaire. Je veux encore une fois remercier l'ensemble des parlementaires qui se sont saisis de cette PPL pour donner corps à la protection du droit à la formation. Je vous remercie.-- Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a introduit une réforme audacieuse du compte personnel de formation qui a permis une démocratisation de l'accès à la formation professionnelle au bénéfice de chaque actif.-- la monétisation du CPF et le lancement du service des des mayas dématérialisé excusez-moi mon compte formation, lui ont donné une nouvelle dimension. Environ 2.100.000 dossiers de formation ont ainsi été financés en 2021, contre près d'un million en 2020 500.000 en 2019, soit un doublement chaque année. Grâce à un mode d'alimentation, favorable au temps partiel. La réforme a également permis un rééquilibrage du recours au CPF entre les hommes et les femmes.-- Les actifs de moins de 40 ans et les publics peu diplômés sont également plus représentées parmi ces bénéficiaires. Toutefois, cette réforme a aussi une face sombre. Avec 19 millions de profils activé sur mon compte formation à a ouvert une brèche dans laquelle divers acteurs peu scrupuleux se sont engouffrés pour se livrer à des pratiques frauduleuses.-- La fraude au CPF prend des formes diverses allant de pratiques commerciales agressives à la validation d'entrer en formation fictive ou inéligible à un financement par le dispositif.-- Les titulaires du de comptes sont selon les cas, victime ou complice de ces abus.-- La Caisse des dépôts et consignations évalue à 40 millions d'euros au Bammou. Le préjudice financier il y a ces pratiques.-- Ce montant reste peu élevé au regard des dépenses totales occasionne occasionnés par le dispositif qui se sont élevés à 2,85 milliards d'euros en 2021.-- La situation pourrait néanmoins s'aggraver en l'absence d'action rapide et ferme pour faire cesser ces agissements. De plus, au-delà de leur impact financier ces pratiques nuisent à l'image du CPF et plus généralement à celles de l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle.-- La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui déposée par les des plutôt député Bruno Fuchs Sylvain Maillard et Thomas Mesnier, état et adopté par l'Assemblée nationale le 6 octobre dernier vise donc à rendre plus efficaces les efforts déployés pour lutter contre ces abus.-- Je salue à cette occasion, Catherine Fabre qui était à l'initiative de la première proposition de loi en ce sens et je la remercie de sa présence parmi nous.-- Depuis le lancement de mon compte formation en novembre 2019, la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle. La direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences et la Caisse des dépôts et consignations gestionnaire du CPF coopèrent en matière de lutte contre la fraude. Leurs efforts se sont amplifiés depuis le 2021 en raison de l'aggravation du phénomène. Ainsi, des mesures fortes ont récemment été prise dans le but de tarir les sources de la fraude.-- Depuis le 25 octobre dernier, afin de prévenir les usurpations d'identité et les utilisations frauduleuses du compte l'accès des utilisateurs à la plateforme a été sécurisé par la mise en place de la solution France Connect plus. En alourdissant le processus de connexion. Cette mesure a eu des effets immédiats. Même s'il convient de veiller à ce qu'elle ne conduise pas à exclure les personnes en difficulté avec le numérique.-- Le volet contentieux de l'action de la Caisse des dépôts commence lui aussi a porté ses fruits avec la première condamnation pour fondre au CPF. Le 20 septembre dernier à Saint Omer d'un organisme qui avait organisé de fausses sessions de formation.-- Il reste néanmoins des obstacles législatifs à lever pour permettre à ces actions de produire leurs effets.-- En matière de démarchage téléphonique. La loi du 17 mars 2014 relatives à la consommation. à la consommation a mis en place un régime d'opposition à travers la possibilité de s'inscrire gratuitement à la liste Bloctel. Ce régime a été renforcée par la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique qui a rendu obligatoire la consultation par les centres d'appels de la liste d'opposition et alourdit les sanctions applicables.-- Pour les courriers électroniques et SMS un régime de consentement préalable et explicite s'applique.-- Ce dispositif n'ont pas empêché la prolifération de pratiques agressives de démarchage relatif au CPF. Le téléphone est le principal vecteur de prise en contact entre les organismes de formation et les titulaires de comptes, mais ce n'est pas le seul.-- Face à ce constat, l'article 1er de la proposition de loi tend à interdire la prospection commerciale des titulaires d'un CPF par téléphone par SMS par courriel ou sur les réseaux sociaux visant à collecter leurs données à caractère personnel ou à conclure des contrats portant sur des actions de formation, sauf si la sollicitation intervient dans le cadre d'une action de formation en cours et présentant un lien Direct avec son objet.-- Afin de contrôler le respect de ces dispositions, il habilite les agents de la DGCCRF. À rechercher et constater ces infractions et prévoit des sanctions administratives d'un montant maximal de 750.000 de 75.000 euros pardon pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. Cette mesure stricte n'empêchera pas les organismes de formation de communiquer mais permettra de faire cesser le démarchage abusif en clarifiant les règles. À l'aura également les actifs à prendre des décisions réfléchies sur l'utilisation de leur CPF et le choix de leur avenir professionnel.-- La proposition de loi vise par ailleurs à renforcer les moyens d'action de la Caisse des dépôts et consignations face à la fraude. À cette fin, elle donne une base légale à la communication d'informations entre les acteurs concernés. L'article 2 prévoit ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les services de l'État chargés de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mais aussi les organismes financeurs. Les organismes délivrant la certification Kaliopie et les ministères ou organismes propre aux propriétaires de certification professionnelles peuvent échanger tous documents et informations détenues ou recueilli recueilli dans le cadre de leurs missions respectives et utile à leur accomplissement. Il autorise également la cellule nationale de renseignement financier Tracfin à transmettre des informations à la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'à l'Agence des services de paiement.-- La sécurisation juridique de ces échanges d'information permettra de faire gagner un temps précieux à la Caisse des dépôts pour l'accomplissement de sa mission de lutte contre la fraude.-- L'article 2 bis inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement donne à la Caisse des dépôts et consignations, les moyens de mettre en oeuvre a recouvrement forcé des sommes indûment en verser à un organisme de formation.-- À cet effet. Le directeur général de la Caisse des dépôts pourra délivrer une contrainte qui à défaut d'opposition du prestataire devant la juridiction compétente. Comportera tous les effets d'un jugement. En outre. Lorsqu'elle constatera la mobilisation par le titulaire d'un CPF de droits indus ou une utilisation contraire à la réglementation. La Caisse des dépôts pourra procéder au recouvrement de l'Hindu par retenue sur les droits inscrits ou sur les droits futurs du titulaire.-- Comme le prévoit l'article de. Les agents de la Caisse des dépôts pour obtenir de l'administration fiscale les informations contenues dans le fichier des comptes bancaire le Ficoba. En outre, la Caisse pourra recevoir de l'administration fiscale communication de tous les documents ou renseignements nécessaires au contrôle préalable au paiement des sommes dues, ainsi qu'à la reprise au recouvrement des sommes indûment indument versées au titre du CPF. L'article 3. À inscrire dans la loi, les conditions du référencement sur mon compte formation, ce qui permettra de fonder le refus par la Caisse des dépôts de référence et un organisme de formation qui ne remplirait pas ses conditions.-- Il serait notamment vérifier que l'organisme propose des formations éligibles à un financement CPF dispose de la certification qualité Kaliopie respectent les prescriptions de la législation fiscale et sociale est satisfait aux conditions générales d'utilisation. La Caisse pourrait procéder à la même vérification pour les organismes de formation déjà référencés sur la plateforme. Avant la publication de la loi. Afin d'assurer l'opérationnalité de la mesure des échanges de données pourraient être organisées entre la Caisse des dépôts et consignations les Urssaf et l'administration fiscale.-- Afin de mettre à certaines enfin à certaines dérives de nature à tromper les titulaires de CPF. L'article IV vise à encadrer le recours à des sous-traitants en soumettant ces derniers aux mêmes obligations que les donneurs d'ordres. Cette dernière mesure appellent une vigilance particulière appliquer indistinctement à tous les sous-traitants notamment les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs, elle pourrait mettre en péril une partie du secteur. Le décret en Conseil d'État prévue pour son application devra bien préciser la portée de ses obligations selon le degré d'implication dans l'exécution des actions de formation et la nature du prestataire concernés. Madame la ministre, nous comptons sur vous pour appliquer ces dispositions avec discernement et bonne Intelligence avec les représentants du secteur de la formation professionnelle et vos propos à l'instant démontre votre volonté aller en ce sens. Mes chers collègues. L'adoption de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale a déjà eu un impact psychologique. Il s'agit aujourd'hui de ne pas laisser cet effet se dissiper. Et de ne pas retarder l'entrée en vigueur de ce texte utiles et attendus. Je vous invite donc au nom de la commission des affaires sociales a adopté sans modification. Cette proposition de loi, je vous remercie. C'est le président, madame la ministre. Mes chers collègues, nos concitoyens subissent depuis des mois des campagnes massives de démarchage téléphonique concernant le compte personnel de formation. Ces appels incessants pour objectif tantôt de s'enquérir du solde de leurs comptes tantôt de les insister lourdement à souscrire à des formations plus ou moins douteuses ou sérieuse. Le compte personnel de formation est un formidable outil au service de nos concitoyens de leur compétence et de leur productivité depuis 2015, il permet aux Français qui le souhaitent de financer des formations continues grâce à leur cotisation que ce soit pour se perfectionner dans leur emploi actuel ou bien pour ce gros convertir dans une autre voie professionnelle, les Français sont, sont largement emparés rançon du succès. À mesure que le nombre de formation continue d'être dispensé. Le nombre de fraudes lui lui s'est multiplié dans le flot des sollicitations que nos concitoyens reçoivent de nombreuses offres ne sont pas légitimes poussé à conclure des contrats de formation, beaucoup ont constaté que la qualité n'était pas au rendez-vous. Puis encore que certaines formations ne sont tout simplement pas dispenser les fraudeurs se contente d'encaisser le paiement. Dans un domaine qui est en train de devenir un véritable Far-West. Il nous faut légiférer. C'est tout l'objet de la proposition de loi portée par notre collègue Martin lévrier voté à l'Assemblée nationale avec le soutien du gouvernement ce texte propose plusieurs mesures de bon sens et pose tout d'abord le principe de l'interdiction de tout démarchage relatif au compte personnel de formation. Il se trouve que ce matin j'étais au téléphone avec un maire, le maire de Nozay qui me disait que tous ces élus sans exception avaient tous été appelé pour être je dirais pousser à une formation qui n'avait pas de sens. Bien entendu, cette interdiction ne s'oppose pas à ce que le bénéficiaire d'une formation souscrites soient contactés par l'organisme. Pour les besoins de cette formation ensuite cette proposition de loi met fin à une pratique problématique à bien des égards le portage quoi lui pouvait s'apparenter à un détournement de certification qualité une société certifié faisait bénéficier une société qui ne était pas de sa certification désormais sous-traitants non les organismes de formation auront l'obligation d'être référencé auprès de la formation de la plateforme mon compte formation, cette obligation est suivi de cette. Le procès de produire des justificatifs attestant le sérieux et la qualité des formations à six dispensés enfin les instances chargées de la lutte contre la fraude voient leur capacité de coopération renforcée en échangeant leurs informations, elles seront plus efficaces dans leur mission. Nos concitoyens ne seront plus importuné auront accès à des formations de qualité, le renforcement du contrôle du système de contrôle du compte personnel de formation permettra de mettre un coup d'arrêt à la fraude qui se développe. Bref, un consensus se dessine autour de ce texte. Nous souhaitons que l'adoption de ce texte équilibré soit la plus rapide possible. Ah si nos concitoyens pourront bénéficier au plus tôt de ses effets. L'ensemble du groupe les indépendants votera donc en faveur de cette excellente proposition de loi

Merci. Merci monsieur le président, madame le Ministre, chers collègues. Les Français et les Françaises il fait froid. Reçoivent en moyenne 5 appels non désirés, chaque semaine, le dernier rapport de traque fine, fait état d'une augmentation des fraudes téléphoniques détecter d'environ 450% en un an. Une hausse qui est grandement due aux fraudes au CPF, c'est évidemment insupportable. Personne ne veut recevoir des appels et des SMS persistant pour la plupart des arnaques et cela à participer à l'émergence d'un consensus transpartisan pour lutter contre ces fraudes. Évidemment que le problème ce sont les arnaques et évidemment que le groupe écologiste votera en faveur de cette proposition. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est l'environnement qui fait prospérer ces arnaques, la monétarisation du CPF son passage d'heures en euros, ainsi que la désintermédiation via mon compte formation ont favorisé le développement d'un marché mal régulé et le montage des fraudes. Contre lesquels nous travaillons aujourd'hui. Les écologistes se sont toujours opposés aux modifications qui produit ce genre d'effets délétères. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut aller un peu plus loin et regardez l'environnement général qui rend les abus possibles. Interdire les fraude et le démarchage abusif sur un sujet à la fois et à chaque fois ne change pas le problème de fond puisque nous continuons à en égréner à chaque fois qu'un nouveau marché se saisissent cette possibilité et les outils proposés par l'État comme Bloctel sont malheureusement peu efficace. En réalité le démarchage téléphonique abusif en général et la forme la plus visible des conséquences de la vente de nos données personnelles et du manque de contrôle de la publicité le RGPD, en vigueur depuis 2018 n'imposent le consentement préalable du citoyen et la citoyenne que pour la prospection commerciale automatisé, c'est-à-dire les courriels mails SMS ou télécopie. Les appels téléphoniques bénéficient donc de cette faille alors même qu'ils peuvent être autant voire beaucoup plus intrusif encore qu'un SMS. Alors que faire. Comme souvent, nous pourrions nous inspirer de nos voisins européens, l'Allemagne, l'Autriche, la Lituanie, la République tchèque. On fait le choix de ce qu'on appelle le Optile. Dont les appels commerciaux, c'est-à-dire que le démarchage commercial par téléphone n'est autorisée que si la personne a explicitement donné son accord. On inverse donc le principe actuel et on épargne des millions de personnes de ces nuisances dans cette lignée je défendrai 2 amendements pour améliorer ce texte dans ce sens afin d'interdire le démarchage téléphonique commercial non consentie dans l'ensemble des domaines de prospection commerciale, pas seulement le CPF. Et pour mettre en place un registre d'autorisation des appels afin d'inverser. Si je puis dire, la charge de la preuve. Je conclurai en rappelant que cette loi de ne va pas nous faire perdre de vue non seulement la nécessaire protection de nos données personnelles mais aussi la nécessaire transformation du droit à la formation dans l'optique d'un monde du travail adapté ou nécessaire tournant écologique, le gouvernement prend un virage antisocial en prévoyant d'allonger la durée de cotisation pour obtenir une retraite décente arabe autant le RSA et cetera. Le mot d'ordre c'est travailler plus précarisées pour obliger chacune et chacun à prendre n'importe quel emploi en être en moins bonne santé. Alors que travailler plus pour toujours produit plus. En pleine catastrophe écologique. Ce n'est pas logique nous écologistes, nous pensons au contraire que la question de l'information doit être un outil pensé au service de la transformation écologique de notre économie. Il faudrait donc un droit à la formation pour se reconvertir qui seraient intégrés au compte de formation au compte professionnel de prévention et tout spécifiquement.-- Pour les métiers en transition, il faudrait aussi que le droit à la formation tiennent compte de l'importance de former des individus tout au long de la vie pas seulement dans une optique de professionnalisation au sens strict du terme mais permettre à chacune et à chacun d'apprendre de s'enrichir de connaissances sur différents sujets d'intérêt général de progresser dans la compréhension du monde, même quand ce n'est pas formellement formellement rattaché à un élément de carrière quantifiable un et tout cela participe à la construction d'une société plus ouverte, plus riche, plus intelligente et dans laquelle je crois il ferait meilleur vivre, je vous remercie.--

La fraude au compte personnel de formation. Le CPF a été fortement augmenté en 2021, le nombre de note transmise à l'autorité judiciaire par Tracfin a été multiplié par 3 en un an. 5 pour le montant total des enjeux financiers correspondants et qui est passé à plus de 43 millions d'euros. Afin de mieux lutter contre ces pratiques commerciales plusieurs initiatives parlementaires ont été prises ces derniers mois, celle dont nous débattons aujourd'hui et qui passe et qui est en passe d'aboutir et c'est une excellente nouvelle, a été déposée par les groupes. MoDem Renaissance et Horizons et elle reprend les dispositions du texte de l'ancienne députée de Gironde Madame Catherine Fabre qui est ce matin en tribune et que je salue. Les 3 auteurs nos collègues députés Bruno fiche Sylvain Maillard et Thomas Mesnier, rappelle à juste titre dans leur exposé des motifs que si les CPAS rencontre un succès remarquables. Celui-ci s'accompagne de pratiques commerciales agressives et parfois abusives visant à pousser les individus à acheter des formations contre leur gré et c'est inacceptable. Ces agissements et nous sommes très nombreux à les subir parfois quasi quotidiennes quotidiennement prennent la forme d'appel de SMS de courriels de la part de centres d'appel ou d'organismes de des À cette occasion sont souvent diffusé des informations erronées sur les droits de la formation de l'individu, mais aussi concernant l'objet réel poursuivi par l'organisme. Le temps de la réguler, rajouter la semaine dernière, la commission des affaires ce sociales du Sénat a adopté à l'unanimité et sans modification. Cette proposition de loi. Cette validation fait donc suite à une autre, celle des députés intervenu début octobre là encore à l'unanimité. Nous devons parvenir à une adepte à une adoption définitive du texte parce que ce phénomène retrait gros traitables qui touche des milliers d'entre nous rend plus que nécessaire, le renforcement des dispositions. C'est pourquoi notre groupe a souhaité l'inscrire dans son espace réservé en cette fin d'année notre rapporteur Martin lévrier qui est intervenu à plusieurs reprises sur ce sujet par le passé là justement rappelé, nous considérons que la lutte contre la fraude et l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle forment un continuum et si ce texte n'exprime n'épuise pas le sujet des ajustements apportés au CPF. C'est une première réponse importante le dispositif que nous nous apprêtons à voter vise tout d'abord à interdire le démarchage téléphonique par SMS courriel des organismes de formation en vue de lutter contre la fraude au CPF. Pour ce faire il a inscrit cette impossibilité dans le code de la consommation d'une part, selon le même dispositif que MaPrimeRénov. Dans le code du travail, d'autre part, dès lors que ce démarchage n'a pas lieu dans le cadre d'une prestation en cours entre un individu et un organisme de formation. Il entend également renforcer les capacités d'action de la Caisse des dépôts en matière de lutte contre les fraudes et en facilitant les possibilités de recouvrement des sommes indûment perçues. Il encadre aussi le recours à la sous-traitance par les organismes de formation. Intervenant sur la plateforme mon compte formation. Sur ce dernier point en réponse à l'inquiétude d'une partie des acteurs du marché de la formation, vous avez alerté le gouvernement. Monsieur le rapporteur. Sur les personnes ayant le statut d'auto-entrepreneur et qui auront toutes les difficultés à rentrer dans les critères de la certification qualité Kaliopie. C'est pourquoi il est prévu que la déclinaison de cette dispositions soient prises par décret permettant ainsi une meilleure adaptation aux spécificités de chacun, si ce texte est adopté sans modification. Alors la promulgation devra intervenir rapidement pour une application dès le début de l'année 2023, nous ne sommes, je le crois très attendu sur ce point, il est de notre devoir de dépolluer les pratiques illégales qui créent un du monde la dépense ternissent l'image du CPF et dépose le titulaire de son libre arbitre, c'est ce que vous avez justement rappelé Madame la Ministre nous voterons pour et je vous remercie.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur. Pour mémoire, le compte personnel de formation a été créé par la loi de réforme de la formation professionnelle à l'emploi et la démocratie sociale. Entré en vigueur en 2015, en remplacement du droit individuel à la formation. L'objet du CPF était de rendre son efficacité à l'appareil de formation professionnelle initialement organisée par la loi de l'or, de 1971. Texte qui a institué la possibilité pour le salarié de bénéficier, à son initiative d'un congé de formation rémunérée il obligeait également les entreprises de plus de 10 salariés à participer au financement des actions de formation. Dans sa continuité. La loi de réforme de la formation professionnelle à l'emploi et à la démocratie sociale votée sous majorité socialiste en 2014, a donc permis de jeter les bases d'une véritable sécurité sociale professionnelle. Elle a en effet mis en place le compte personnel d'activité qui regroupe les droits du salarié, avec le compte personnel de formation. Le compte de prévention de la pénibilité et le compte engagement citoyen. On sait le sort réservé par l'actuel gouvernement à ses acquis sociaux alors que nous avions par la loi de 2014. Renforcer la place des partenaires sociaux, en faisant de la formation professionnelle, un élément central du dialogue social, nous rappelions également notre attachement au mouvement de décentralisation de la formation professionnelle, vers les régions. En 2018, lors des discussions engagées ici même sur le projet de loi. Liberté de choisir son avenir professionnel. Nous dénoncions un texte qui allait fragiliser l'édifice que nous avions construit le projet de loi présenté par la ministre du Travail d'alors, devait en effet prétendument en être un volet sécurité des transitions professionnelles en contrepartie des ordonnances travail visant à fluidifier le marché du travail auquel nous étions et De Meuron foncièrement opposé en tout état de cause, le compte n'y était pas. Nous n'avons pu que constater que c'est la première réforme de la formation professionnelle qui ne faisait pas consensus. Depuis 1971, elle a abouti à une véritable recentralisation. Dans une logique qui porte la marque de fabrique de l'actuel président de la République et de ses ministres, le gouvernement s'est en effet assis sur la démocratie sociale en instaurant la monétisation du compte personnel de formation en dépit du rejet unanime par les partenaires sociaux de cette évolution en monétisent en le CPF en supprimant les intermédiaires et un imposant le recours à une plateforme numérique la majorité disait vouloir libérer les salariés et leur offrir plus de droits. Nous nous inquiétons qui ont, quant à la pérennité du financement du CPF et des risques induits par la désintermédiation et la monétisation. Il semble que nous ayons eu raison. Concernant les enjeux du financement dans le rapport d'information relatif à France compétences publié en juin 2029 par 4 sénateurs dont notre collègue Corinne Ferré co-, rapporteur de la mission à l'origine de ce document, il est en tout état de cause signaler que les besoins de financement n'ont pas été anticipée, France compétences établissement public chargé du financement et de la régulation de la formation professionnelle pourrait afficher un déficit de 5 milliards 900 millions d'euros en 2022. Le problème de la fraude au CPF qui est le sujet de la présente, proposition de loi était également en germe dans la loi de 2018, le résultat on le connaît. Entre le 1er semestre 2021 et le premier semestre 2022, les signalements de SMS indésirables ont été multipliés par 14. Les déclarations de soupçons liées à une potentielle fraudes au CPF ont été au CPF ont été multipliés par 11, 32.400 signalements ont été effectués auprès de la Caisse des dépôts, gestionnaire du dispositif au 1er semestre 2022. Le préjudice estimé dans le cadre des plaintes pénales déposées par la Caisse des dépôts, entre mars 2020 et mai 2022 s'élève à 27 millions d'euros les fraudes détectés par Tracfin sont passés de 8 millions d'euros en 2020 à 43 millions d'euros en 2021 soit une augmentation de l'ordre de 450%. Les propositions portées par la présente, proposition de loi sont nécessaires et consensuel et nous y souscrivons bien sûr elle interdit à l'article 1 toute prospection commerciale des titulaires d'un CPF par voie téléphonique par SMS mais aussi par courrier électronique ou en ligne sur un service de réseaux sociaux. Dans le but de permettre le contrôle effectif de l'interdiction du démarchage et titulaire du CPF. Elle prévoit à l'article de d'étendre les pouvoirs des agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes afin que ces derniers soient habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements à cette interdiction. L'article 2 bis introduit par le gouvernement en séance à l'Assemblée nationale mais de nouveaux outils à disposition de la CDC pour faciliter le recouvrement des fonds versés de manière indue ou suite à une fraude du titulaire du CPF. L'article 3 de la proposition de loi prévoit d'introduire d'imposer aux organismes de formation d'adresser à la Caisse des dépôts, une demande de référencement sur la plateforme mon compte formation. L'article 4 également introduit par le gouvernement en séance à l'Assemblée prévoit enfin d'certaines des obligations liées au référencement des organismes de formation sur la plateforme mon compte formation ou sous-traitants. Actuellement, lorsqu'un organisme de formation a recours à un sous-traitant pour effectuer les actions de formation proposée sur son catalogue. Ce dernier n'est pas soumis aux conditions générales d'utilisation. C'est nécessaire correction nous y souscrivons mais tout comme le pays nous sommes fatigués de naviguer, d'usine agace en usine agace le démantèlement de la démocratie sociale par le gouvernement et ses choix dommageable en termes de droit du travail ayant des conséquences que nous ne faisons que commencer à réparer. Sur ce texte bien particulier. Notre groupe votera favorablement.-- Merci, cher collègue, la parole est ensuite à Madame Katia pour polie pour le groupe CRCE. Et pour quatre minutes à nouveau.

et d'interdire le démarchage de 6 titulaires, a été adopté à l'unanimité le 6 octobre 2022 à l'Assemblée nationale en première lecture. Elle vise à mettre fin aux des marchands démarchage incessant et intempestifs émanant d'organismes pour certains fictif. La création du compte personnel de formation, couplé à la monétisation des heures de formation ont entraîné l'émergence d'un démarchage agressif avec son lot de fraude. Pas un jour ne passe sans que son lot de SMS d'appel ou de mail invitant à utiliser son crédit du CPF. Cette situation insupportable pour nos concitoyens était possible, avec évidemment la transformation des heures de formation en 2018 en montant financier a utilisé par la loi Pénicaud. Il est d'ailleurs difficilement acceptable que l'ex-ministre du travail, à l'origine du Big bang de la formation professionnelle de 2018 s'apprête à entrer dans le conseil d'administration de Galiléo Global Éducation un énorme groupe d'enseignement supérieur privé acteur majeur de la formation initiale et continue. En attendant l'interdiction de la prospection commerciale des titulaires d'un compte. Personnel de formation assorti de sanctions pour les entreprises non respectueuses de cette interdiction est une bonne nouvelle. Il est regrettable qu'il ait fallu attendre 4 ans pour étendre. S'attaquer à ce fléau et a doté de prérogatives de contrôle des agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. La montée en puissance du CPF s'est accompagnée d'une hausse massive des fraudes et des tentatives de fraude entre 2020 et 2021. Ça été rappelé le nombre de déclarations de soupçons liées à une fraude potentielle au CPF a été multiplié par 11 et celui des dossiers transmis à la justice par Tracfin sur ce thème par trois d'un côté nous avons des organismes fictifs qui ont des pratiques frauduleuses et de l'autre des organismes réel qui effectue du démarchage agressif. L'eau probe est jetée sur l'ensemble des organismes de formation y compris ceux qui ne sont pas dans l'illégalité. Espérons que le référencement des organismes de formation sur le portail numérique mon compte formation permettra de faire le tri entre les organismes sérieux et les autres. Je voudrais profiter de ce texte pour alerter sur la présence d'organismes de formation aux pratiques sectaires qui piège les salariés qui utilisent leur compte de formation. Le dernier rapport d'activité de Milly MIVILUDES fait état d'une augmentation globale des dérives sectaires, avec un record de 4020 saisines en 2021 et 86% d'augmentation entre 2015 et 2021. La formation de coaching de techniques de vente de développement personnel ou de techniques de soins non reconnue font l'objet d'un nombre très important de signalement. Il faut donc renforcer la formation permanente des agents chargés du contrôle face à ces dérives. Enfin je voudrais signaler que l'examen de cette proposition de loi se fait dans un contexte de restriction de la lie de l'accès à la formation professionnelle avec l'instauration d'un reste à charge par le gouvernement. Le projet de loi de finances pour 2023 que nous avons adopté mardi prévoit de contraindre les salariés à prendre en charge, 20 à 30% du coût de la formation. Cette remise en cause du droit à la formation qui pénalisera en 1er lieu les salariés les plus modestes et les privés d'emploi est évidemment inacceptable. Nous défendons une formation professionnelle accessible tout au long de la vie aux travailleurs et aux privés d'emploi, intégralement financés par les entreprises. En attendant, notre groupe votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur le président, madame la ministre madame la rapporteure, mes chers collègues. la loi du 5 septembre 2018 intitulé pour la liberté de choisir son avenir professionnel à réformer le compte professionnel de formation créée en 2014, le principe de droit en heure a été transformé, remplacé par un dispositif monétiser en euros en allant sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Des chiffres, il s'affiche en gros caractères, nombre de personnes titulaires d'un compte CPF au 30 septembre 2021. 38,8 millions. Montant moyen par CPF. 1500 euros. Nombre de dossiers acceptés entre novembre 2019 et le 30 septembre 2021 de. 86 millions n'importe quel malfaisant. Pas très malin a vite fait de comprendre avec une soustraction une multiplication qu'environ 36 millions de salariés n'ont pas mobilisé chacun leur 1500 euros de CPF et qu'il y a là une gigantesque arnaque à mettre en place ce qui n'a pas manqué. Et ce sont même des malfaisants très malin qui ont sauté sur l'aubaine. Les premières fraudes fut relativement simple proposant de fausses formation et usant de fausses identités. Malgré le renforcement des dispositifs de contrôle Tracfin constaté en 2021 une persistance voire un renforcement de la fraude qui s'organisent au fur et à mesure de la tentative de sécurisation du dispositif. Désormais, on constate des inscriptions fictives à des formations non suivi un démarchage agressif et même des incitations d'inscription par des offres de cadeaux. Derrière ces pratiques, il y a des réseaux de criminalité organisée dont des affairistes, déjà connu, dans le cadre de fraude aux certificats d'énergie qui ont mis la main sur le dispositif plusieurs dossiers ont donné lieu à des saisies pénales effectives pour un total de 3, 5 millions d'euros. Parmi les dossiers, les 20 dossiers transmis 10 mettent au jour des réseaux de fraudeurs particulièrement structuré et rattaché à des groupes criminels organisés. Voici un exemple réel la société spécialisée dans l'information continue d'adultes et dirigé par Monsieur X créé en septembre 2020 ne déclare aucun salarié elle reçoit plus de 8 millions d'euros de la Caisse des dépôts et consignations au titre du CPF sur la base de fausses attestations de stagiaires. Une part importante des sommes perçues par la société a aussi du CPF et transféré vers des personnes physiques et morales liées à Monsieur X dont des sociétés actives dans les secteurs du BTP du Conseil pour un million d'euros, une association présidée par le frère de Monsieur X 3 millions d'euros et de membres de la famille de Monsieur X 200.000 euros une partie des fonds versés sur le compte de l'association est utilisée pour l'achat de véhicules et de montres de luxe par le frère de Monsieur X, enfin 300.000 euros perçus par la société à au titre du CPF ont été transférés en faveur de personnes physiques enregistré comme stagiaire de la société ayant initialement sollicité le paiement du CPF. Au cours de l'année 2021, la Caisse des dépôts a procédé à l'arrêt des versements à la société a otite du CPF en raison de graves soupçons de fraude. Ce sont finalement plus de 2 millions d'avoir qui ont pu être saisis et confisqués qu'par l'Agrasc mais 6 millions qui se sont potentiellement évadé. C'est pourquoi sans hésiter sans état d'âme et afin que ces pratiques de démarchage sont rendues impossibles dans les meilleurs délais, nous voterons en l'état le texte qui nous proposée aujourd'hui. Il faut que cela cesse au plus vite et pas en mettant en place des procédures dématérialisées plus complexe mais en réussissant finalement à bloquer l'accès aux numéros des bénéficiaires. En effet, ce ne sont pas les personnes déjà éloignés du numérique, il faut écarter mais bien les bandits financier face à ce constat de fraude exponentielle. L'article 1er de ce texte de loi tend à interdire la prospection commerciale des titulaires de comptes formation sauf sollicitations explicite dans le cas d'une forme d'actions de formation en cours. C'est très bien mais la vraie question qui se pose en fait, c'est de savoir comment les acteurs du grand banditisme ont libre accès à ces fichiers face à la circulation de toutes nos informations personnelles dans tout l'éclat ou du monde reste-t-il une possibilité de verrouillage car faut d'agir sur la sécurité des fichiers après s'être fait arnaquer hier sur les deux dossiers d'isolation aujourd'hui sur les dossiers de formation. L'État et les citoyens se font arnaquer demain sur d'autres dossiers et ce sera toujours plus juteux plus organisée, plus efficace et de plus grande ampleur. L'article de prendre le contrôle par l'échange et le croisement d'informations entre les services, ce qui semble de pur bon sens et même élémentaire. C'est du fonctionnement des services en silos que naisse et prospère toutes les supercheries les plus énormes. Il semble que les outils informatiques auraient dû permettre depuis longtemps le recoupement systématique des données et dans dans tant de Nomen. Ce serait donc à généraliser. Près, vous aurez compris que l'ensemble de ces lois va dans le bon sens mais toujours hélas a posteriori, une fois que l'on est débordé et que le Torrent semble si difficile à contenir. Je pose à cette occasion, la question des moyens du contrôle et de son coût et j'espère que tout est calibré à hauteur de l'enjeu mais ne répondait pas ici car des oreilles malhonnête pourrait, écoutez. Je voudrais conclure en rappelant les débats que nous avions il y a eu quelques mois au sujet d'une proposition législative d'interdire complètement le démarchage téléphonique en général. Nous avions alors rappelé le dispositif Bloctel qui permet théoriquement de se protéger et nous avions décidé de surseoir à cette décision afin de respecter des milliers d'emplois de salariés honnête. Nous sommes aujourd'hui dans un autre cas de figure, l'interdiction du démarchage compte CPF ne contrariera que des opérations frauduleuses. Alors allons-y, je vous remercie.

Monsieur le président. Monsieur. Monsieur le. Le rapporteur. Chers collègues. Le compte personnel de formation a fait l'objet d'une réforme en 2018 dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L'objectif que nous partagions était de rendre les droits à la formation plus lisibles plus accessibles en créant notamment une plateforme internet sur laquelle chaque personne pourrait connaître le montant de ces droits désormais visibles en euros choisir et payer directement sa formation sans intermédiation. Lancé fin 2019. Mon compte formation a permis l'activation de 19 millions de profil et l'augmentation très nette du nombre d'entrants en formation dans toutes les catégories professionnelles et c'est à souligner les femmes notamment plus souvent à temps partiel, bénéficient de l'alignement des droits, avec un compte alimenté de 500 euros par an pour tous les salariés qui effectuent au moins à mi-temps et 800 euros pour les moins qualifiés ou en situation de handicap. Cette réforme que nous jugions et que nous jugions et jugeons souhaitable à l'époque et dont nous constatons aujourd'hui. Le succès a rendu les Français plus libre d'évoluer professionnellement. Et nous savons à quel point la question de la formation est central dans la recherche de l'adéquation entre les profils des demandeurs d'emploi et les offres du marché du travail. Mais tout changement entraîne des effets de bord. Nous sommes en plein dans la montée en puissance du CPF s'est en effet accompagnée d'une hausse massive des fraudes, des tentatives de fraude ainsi que d'un harcèlement pour appels téléphoniques, SMS courriels démarchage sur les réseaux sociaux. Cela a été évoqué par les orateurs précédents, le phénomène a pris une ampleur considérable depuis plusieurs mois et je crois que nous pouvons tous le confirmer pour certains d'entre nous l'avoir subi au-delà des pratiques commerciales agressives abusive les informations erronées sont véhiculées induisant en erreur les titulaires des comptes ou en les poussant à acheter des formations contre leur gré. C'est aujourd'hui une nuisance réelle qui a envahi le quotidien des Français et qui met en péril la crédibilité du dispositif et du secteur de la formation professionnelle. Tracfin. Évalue la fraude à 43 millions d'euros en 2021, nous devons effectivement y mettre un terme au plus vite cette proposition de loi nécessaire et bienvenu vise à rappeler que le CPF est un outil destiné à ceux qui le détiennent et non aux organismes de formation. Les Français doivent impérativement garder la main sur leurs droits. Les dispositifs mis en place jusqu'ici pour contrôler la qualité des formations et sanctionner les manquements et les fraudes n'ont malheureusement pas permis de lever toutes les difficultés. Il s'agit donc de mettre en place des barrages filtrants, rendant plus compliqué les contournements. À défaut de pouvoir totalement les supprimer 5 solutions concrètes sont ainsi proposés, premièrement l'interdiction avec amende dissuasive. Vous l'avez dit Madame la Ministre de toute prospection commerciale visant les titulaires d'un CPF. À l'exception des sollicitations qui interviendrait dans le cadre de prestations en cours. Deuxièmement, la sécurisation de l'échange d'informations entre les acteurs mobilisés dans la lutte contre la fraude au CPF, troisièmement le renforcement des pouvoirs de recouvrement des indus de la Caisse des des Quatrièmement, le renforcement des modalités de contrôle du référencement des organismes de formation sur mon compte formation et enfin l'encadrement du recours à la sous-traitance des organismes de formation qui imposera aux sous-traitants les mêmes exigences et donnera à la Caisse des dépôts, les moyens de contrôle de vérification et d'intervention nécessaires. Des ajustements sont nécessaires et les solutions proposées ici semblent consensuel. Cette proposition de loi a été adoptée il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale si nous l'adoptons notre tour sans modification. Et nous avons entendu le message, elle pourra s'appliquer sans délai pour cette raison pour que ces nuisances cessent au plus vite. Notre groupe RDSE votera en faveur de ce texte sans modification. Merci cher collègue. Et enfin Madame Dominique Estrosi Sassone. Pour les républicains. En plus la discussion générale pour huit minutes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur. Mes chars collègue utilisable par tous, tout au long de la vie active, y compris en période de chômage. Le compte personnel de formation, et au moins un succès quantitatif, avec un doublement des effectifs chaque année 500.000 formations demandé en 2019 plus d'un million en 2020 et plus de 2 millions en 2021. Toutefois, si la monétisation du CPF a favoriser sa démocratisation. Elle a également eu des effets pervers avec une fraude en tous genres et des démarchages abusifs dans le sillage du CPF un lot de pratiques douteuses incontrôlables et incontrôlées sont apparus, usurpation d'identité et détournement des droits nuisances par des appels et sollicitations intempestives. Le CPF qui pèse pour 2 7 milliards d'euros de dépenses, soit un 5ème du budget de France compétences attire désormais une délinquance économique organisé comme le démontrent des 45 des Enquête ouverte par le Service central du renseignement criminel de la gendarmerie. La recrudescence atteint même des sommets puisque selon la cellule de renseignement Tracfin 2021 a été marqué par la plus forte hausse de faux organisme détecté avec un préjudice cumulée de 43, 2 millions d'euros après démarchage téléphonique ou en ligne, soit une multiplication par six de la fraude en seulement un an. Force est donc de constater que le récent guide de prévention contre les arnaques publié par le ministère de l'Économie et des Finances n'aura pas été efficace ni les timides campagnes de sensibilisation. L'action du Parlement et donc pleinement nécessaires pour endiguer ce phénomène. Pourtant dès 2018, le Sénat avait mis en garde et exprimé des réserves sur la monétisation et la désintermédiation du CPF. Le gouvernement avait déclaré qu'il s'agissait d'un Paris s'il a permis à un plus large public d'accéder à la formation, il a occasionné des dérives que l'on s'efforce désormais de traiter avec ce texte. Cette proposition de loi est donc la bienvenue afin de contrer des pratiques qui siphonne des crédits destinés à la formation professionnelle. Un programme déjà difficilement pilotable compte tenu des rallonges budgétaires répétées et voter en France compétences en loi de finances. Le CPF n'a pas, par conséquent, pas un seul euro à perdre. Face à la fraude. Les pouvoirs publics ne sont pourtant pas rester inactif. Je tiens à saluer plus particulièrement le travail des forces de l'ordre qui, grâce à des enquêtes minutieuses et complexe ont réussi à démanteler plusieurs réseaux de faux organismes cours des dernières semaines, dont un dans les Alpes-Maritimes à Cannes, Mandelieu où le préjudice s'élever à 8. 2 millions d'euros. Cette proposition de loi permettra non seulement d'en finir avec ces escroqueries mais aussi de restaurer l'image dégradée du du CPF qui, faute de réponses adaptée perd en visibilité. En effet, bon nombre de Français ne prennent plus les appels ou textos au sérieux avec le risque de se détourner de leur CPF pourtant essentiel au cours de leur carrière professionnelle à l'avenir. La question du financement des formations sera aussi un enjeu de nature à réduire la fraude tout particulièrement contre celle qui est consenti par des actifs dans le cadre de la revente des codes d'accès CPF. Comme l'a proposé et voté le Sénat le 28 novembre dernier dans le cadre de la mission Travail et emploi du projet de loi de finances pour 2023, instaurer un plafonnement de prise en charge par le CPF du coup de certaines formations seraient de nature à sécuriser le CPF, au travers d'un mécanisme de régulation j'espère ainsi que l'amendement adopté au Sénat accueillie avec un avis de sagesse du gouvernement. Obtiendra votre soutien. Madame la ministre. Une fois le 49.3 de nouveau dégainé à l'Assemblée nationale, ce qui est vrai pour le budget de la Sécurité sociale l'aussi pour la formation, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Si nous voulons que les salariés participent plus activement à la lutte contre la fraude mais aussi à leur parcours professionnel, sans se contenter de répondre à un appel ou un message leur signalant qu'ils ont du crédit sur leur CPF. Il faudra en passer par un texte par un reste à charge encadrés sans pour autant en faire une barrière tarifaire cette piste avait d'ailleurs été mises en lumière par l'excellent rapport de Madame, Frédérique Puissat Corinne Ferré et de vous-. Même monsieur le rapporteur. Enfin en matière de prévention contre la fraude. L'arsenal de la Caisse des dépôts contient les conditions générales d'utilisation auquel doivent se conformer les 44.000 organismes de formation dont certaines Start-Up innovantes essentiellement digitale plusieurs de ces organismes qui ont dynamisé le secteur m'ont fait part de la rigidité dans la mise à jour des conditions générales d'utilisation et de délai très court pour six. Avec un risque juridique contractuelle pour les formations proposées ne relevant pas du domaine de la loi, je n'ai finalement pas déposé d'amendement visant à laisser un délai minimum de mise à jour des conditions générales d'utilisation aux organismes mais je tiens Madame la Ministre à vous signaler que bon nombre d'entre eux sont inquiets. De l'aveu même du rapport de la commission des affaires sociales, les conditions générales d'utilisation des CGU ont été modifiée à plusieurs reprises, mais la mise à jour demande un important travail juridique qui ne sont pas tous en mesure de fournir, puisque ce n'est pas leur coeur de métier. À ce titre, l'article 3 inscrit dans la loi, les conditions du renforcement des formations sur mon compte formation et établit un contrôle des formations éligibles au financement CPF, au travers de la certification qualité Kaliopie de la législation fiscale de la sécurité sociale mais aussi de la satisfait Satisfaction pardon aux CGU établi par la Caisse des dépôts et consignations. Pourriez-vous Madame la Ministre les renseigner sur ce point précis, il serait en effet regrettable qu'un excès de règles contraignantes succède à un excès de simplification et il souhaiterait ces organismes que la Caisse des dépôts puisse face faire preuve de beaucoup plus de souplesse pour autant. En conclusion, le groupe Les Républicains votera ce texte en l'état et les dispositifs qui sont proposés, qui permettent effectivement de rendre plus efficaces les efforts déployés pour lutter contre les abus de fraudes au CPF. Je vous remercie.

Merci monsieur le président, madame la ministre, chers collègues. Oui merci. Juste une petite intervention comme je l'ai fait la, la semaine dernière en en commission. Monsieur le rapporteur. Ce texte, c'est une avancée importante hein contre pour lutter contre les arnaques constatés autour du compte. Professionnel de, de formation et j'ai bien compris, comme nombre d'entre nous l'importance d'adopter ce ce texte conforme, c'est pour ça que j'ai pas déposé d'amendement. Néanmoins. Le démarchage abusif autour du du peut aussi concerner non non pas seulement le téléphone. Les réseaux sociaux mais aussi les plateformes les plateformes internet à travers de de possibilités. Les publicités entre les vidéos et à l'intérieur des vidéos elles-mêmes pour lesquels on a parfois de la promotion de de formation. Qui pourrait être fini. Avec le compte professionnel de le compte personnel de formation. À travers des influenceurs faisant croire qu'avec telle formation. Vous allez devenir un expert en en placements financiers. Gagner beaucoup d'argent derrière je je caricature un peu mais ça existe. Voilà donc je voulais juste alerter cette proposition de loi et bienvenue évidemment. C'est pour ça que j'ai pas déposé d'amendement et que je la voterai comme l'ensemble de mon groupe. Mais je voudrais pas qu'il y a des failles dans le texte et en tout cas la même liste je demande en tout cas je souhaite que nous soyons même après le vote de ce texte, même après les décrets d'application qui iront. Très vigilant pour pas que s'il y avait des failles ou des trous dans la raquette. Hé bien que certains escrocs si si profite de cette brèche. Voilà je vous remercie. Merci madame la ministre, hein. Une observation.-- Merci monsieur le président, madame la sénatrice, nous partageons cette conviction. Et sa détermination à lutter contre ce type de dérives également. Je voudrais rappeler ce que je disais en en discussion générale il y a quelques instants, l'action qui a déjà été menée par notre opérateur la Caisse des dépôts et des consignations pour adresser des mises en demeure par voie d'avocat. À ses interlocuteurs et est déjà un bon nombre d'entre eux y ont répondu. Comme je disais tout à l'heure autour de 3 axes le 1er c'est l'arrêt de toute publicité en lien avec le CPF qui a déjà été constaté assez largement la mise à disposition de documents. Des sociétés avec qui il était en lien afin de poursuivre des enquêtes et effectuées le le cas échéant, des dépôts de plainte et la troisième c'est au fond un message qui a été diffusé par un certain nombre d'entre eux un message rectificatif. Sur leurs réseaux sociaux pratique et de et de du de de de de la presqu'île égalité finalement de la pratique, la Caisse des dépôts et des consignations a également mené plusieurs actions pour faire cesser ces pratiques commerciales trompeuses. Déjà elle s'est rapprochée de Meta pour tenter d'obtenir non seulement la suppression a posteriori des publications dont, à la connaissance, mais aussi la mise en place d'un mécanisme de filtrage a priori des contenus illégaux. Et d'autre part, la Caisse des dépôts s'est rapproché des grandes agences d'influenceurs pour les alerter sur le sujet. Cette démarche a eu un effet positif puisque les influenceurs de ces agences ont diffusé dès dimanche 13 novembre un message attirant l'attention des followers sur les arnaques au CPF. Évidemment nous poursuivrons les échanges avec ses acteurs, parce que nous sommes comme vous convaincue qu'il faut absolument que ce type de pratiques cessent. Et nous chercherons à poursuivent travaux avec Meta France pour la fermeture des comptes complets, proposant des offres illicites. Voilà, je voudrais vous rappeler que demain nous le gouvernement travaillera aussi avec ses acteurs pour renforcer la la le partage autour de notre détermination à lutter contre ce type d'usage. Merci.-- Monsieur K. Dick demande également la parole sur l'Arctique. Ensuite nous allons voter l'article 1er. Merci parce que ça allait dans le même sens que l'intervention précédente, cette proposition de loi destinée à lutter contre les fraudes au compte personnel de formation est très attendu car elle porte sur un sujet d'une actualité accrue et qui a pris une dimension internationale. J'ai été sensibilisé un aspect particulier de ces escroqueries par un conseiller des Français établis aux Émirats Arabes Unis qui m'a recommandé de prendre attache avec madame Christelle Coiffier que je tiens à saluer ici pour son à une action de lanceuse d'alerte conseillère à l'emploi, Pôle emploi en lien avec la Caisse des dépôts et consignations. Elle s'est rendue compte de ce que font certains influenceurs partie à Dubaï pour tirer parti profit de l'image positive de cet émirat afin de littéralement vendre du rêve de l'argent facilement gagné du soleil toute l'année. Il représente un modèle pour beaucoup, ce qui leur permet de faire la promotion de formation bidon. Certains font même la promotion de formation éphémère pour devenir influenceurs. Confrontés à la détresse de chercheurs d'emploi dans le crédit de formations était épuisé. À force d'avoir couru après 6 Mirage. Madame Coiffier a décidé d'alerter sur son temps libre sur les arnaques au CPF monté par ces influenceurs et a reçu le soutien du Stéphane Vojetta, députée de la 5e circonscription des Français de l'étranger. La proposition de loi qui nous est présenté doit être accompagné d'une prise de conscience de cette dimension internationale car elle va malheureusement de Pair avec l'impunité des escrocs Bruno Lemaire qui a souvent mis en garde les influenceurs sur leurs modes opératoires, a annoncé une table ronde dans quelques jours pour réguler ces pratiques. Cela va dans le bon sens, tout comme cette initiative parlementaire que je soutiens, mais je voudrais vraiment attirer ce l'attention sur cette dimension. à prendre en compte. Merci.-- Merci, chers collègues, je mets aux voix l'article 1er dans la version de la commission qui n'a pas été modifiée qui est pour.-- Abstention il est adopté après l'article 1er, nous avons deux amendements portant article article additionnel qui sont proposées par Madame Vogel, qui a la parole pour le Merci monsieur le président. Écoutez ce premier à un moment, il est assez simple, il consiste à compléter le dispositif pour instaurer le principe général d'interdiction de démarchage téléphonique commercial non consentie en général le 24 juillet 2020 on a interdit les marcheurs téléphonique pour l'isolation des logements et des travaux d'installation de production des Hunger renouvelable, c'est très bien. Un an plus tard, on l'a interdit pour les distributeurs d'assurance en réalité le démarchage commercial non consentie. Ça sous tout le monde, quelles que soient les sujets, donc on propose simplement de l'interdire en général.-- le suivant. En fait il consiste, aujourd'hui on a un mécanisme ou dans une présomption. De consentement au démarchage commercial et on peut s'inscrire sur une liste pour refuser le démarchage. L'idée c'est de passer à une logique inverse d'avoir une présomption de non-consentement au démarchage commercial et de laisser aux aux personnes la possibilité de s'inscrire dans un registre en disant je suis d'accord pour recevoir du démarchage et si les personnes n'ont pas fait ça, hé bien par définition, elles ne peuvent pas recevoir de démarchage et donc inverser la logique, plusieurs pays européens l'ont fait, c'est ce qu'on appelle l'opting ça marche bien et ça soulage des millions de personnes. Merci.-- Donc la Commission va donner son avis sur les deux amendements successivement puis le gouvernement.-- Merci monsieur le président. Ces deux amendements effectivement concerne l'encadrement légal du démarchage téléphonique en général. En conséquence, leur portée dépasse de très loin le simple au sujet du CPF que nous étudions aujourd'hui ces amendements entendent remplacer l'actuel régime d'opposition au démarchage téléphonique, vous l'avez dit matérialisée par le dispositif tel Bloctel pardon, par un régime d'autorisation préalable. L'amendement numéro un en particulier prévoit qu'un professionnel doit avoir obtenu le consentement Express du prospect avant de pouvoir le démarché par téléphone. Quant à l'amendement numéro 2. Il prévoit que seuls sont autorisés les sollicitations effectuées auprès des personnes inscrites sur la liste d'autorisation du démarchage téléphonique. Je rappelle que l'encadrement du démarchage téléphonique a déjà été renforcée. Il y a 2 ans par la loi du 24 juillet 2020. Cette loi a complété le régime d'opposition au démarchage téléphonique en imposant notamment aux professionnels qui contacte un consommateur par téléphone de lui indiquer qu'il peut s'inscrit gratuitement. Avant toute opération de démarchage téléphonique. L'entreprise doit s'assurer auprès de Bloctel que les consommateurs qu'elle entend prospecter ne sont pas inscrits sur la liste d'opposition. La loi a ainsi alourdi les sanctions applicables en cas d'abus. En outre, certaines dispositions de cette loi, ne sont pas encore entrée en application, comme la limitation du démarchage téléphonique à certaines plages horaires. Je propose donc nous en tenir à un dispositif ciblé sur le démarchage au CPF qui pourra ainsi rentrer en application immédiatement. Il conviendra de faire le moment venu un bilan plus général des effets de la loi de 2020, afin de lui rapporte d'apporter d'éventuelles modifications. En conséquence la Commission à un ami a émis un avis défavorable sur les deux amendements.-- L'avis du gouvernement. Madame le Ministre.-- Sont-ils maintenus.-- Bien. Je mets aux voix l'amendement numéro 1 de madame Vogel avec un double avis défavorable qui est pour.-- Qui est contre. Il s'abstient. Il n'est pas adopté, je consulte sur l'amendement numéro 2 est le même vote même vote même. Est pas adopté non plus je mets donc aux voix l'article de non modifié, qui est pour l'article 2. Autre. Abstention il est adopté. Article 2 bis qui. Pour. Contre. À deux abstentions, il est adopté. Article 3 même vote.

Insistant sur le fait que nous souhaitons conclure cette niche avant la coupure du déjeuner que donc la concision des uns et des autres. Serait bienvenue. Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et ternir dire le démarchage de ses titulaires qui est pour.

Avant la bascule sur le second sujet à l'ordre du jour. La parole est à monsieur d'Arnaud pour une mise au point relative un vote vous avez la parole. Le. Oui, merci Monsieur le Président, c'est simplement pour une rectification de vote sur les scrutins publics 95 et 96 où je souhaitais m'abstenir merci.-- Acte est donné de votre mise au point qui sera publiée au JO et figurera dans la veille du scrutin. Je suspends quelques instants pour permettre à chacun et notamment à la ministre. De s'installer pour l'examen du projet du projet point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

Collègues, nous pouvons reprendre la séance.-- L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi. Tendant à la création de délégation parlementaire aux droits de l'enfant. Proposition présentée par monsieur Xavier il a comédie et plusieurs de ses collègues. C'est une demande d'inscription du groupe RDPI. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Xavier Iacovelli, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues. Au moment où nous débutons l'examen de cette proposition de loi visant à créer dans notre assemblée une délégation aux droits de l'enfant. Je reconnais bien volontiers une certaine émotion. Une certaine émotion aussi car pendant longtemps, nous avons cessé collectivement de voir les enfants comme des sujets de droit à part entière. Nous refusons d'admettre que les problématiques, il est touché a été diverse et angles finalement l'ensemble de nos politiques publiques. Une certaine émotion enfin car je sais que cette délégation aux droits de l'enfant est attendu depuis de longs de longue date. Plus de 20 ans par l'ensemble des acteurs à cet égard, permettez-moi de remercier les associations, collectifs et toutes les personnalités engagées qui nous regardent aujourd'hui et qui oeuvrent sans relâche pour que le droit de l'enfant soit davantage reconnue davantage protégés et qui publiquement, on fait le choix de soutenir cette proposition de loi. Le constat est simple, de nombreux défis doivent être relevés pour assurer le respect des droits de l'enfant.-- Si je me félicite de la récente. Création d'une délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale, il n'est pas question ici de jouer le mimétisme.-- Depuis 2018, avec un certain nombre d'entre vous sur tous les bancs, nous avions décidé la création d'un groupe informel pour travailler sur la question de la protection de l'enfance parce que le Sénat se devait d'avoir une entité dédiée aux questions de l'enfance. J'avais également demandé en 2020 la création d'un groupe d'étude au sein de la commission des affaires sociales auprès de sa présidente, mais malheureusement une nouvelle fois, nous avons essuyé un refus. Soyons tout à fait honnête. Cette détermination à travailler sur les questions de l'enfance ne date pas de cette proposition de loi déjà, en février 2003, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi à l'unanimité tant à la création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant présenté par le président du groupe UMP de l'époque Jacques Barrot ce texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat en 2009. Notre collègue du groupe LR Joël Garrigue. Avait déposé cette même proposition de création délégation aux droits de l'enfant au Sénat. Notre rapporteur général du budget de la Sécurité sociale. Élisabeth Doineau avait également proposé la création de cette délégation plus récemment la présidente Assassi et le groupe CRCE ont déposé en 2019 la création d'une telle délégation, vous le voyez, chers collègues, la question de l'enfance rassemble au-delà de nos étiquettes et traverse même le temps. Le texte que je vous présente aujourd'hui le démontre une fois encore car il est assez rare de le souligner que cette proposition de loi est aujourd'hui co- signé par plusieurs sénatrice plusieurs sénateurs de tous les groupes DLR oh CRCE en passant par RDSE centristes, écologistes et socialistes toutes les sensibilités notre chambre y sont représentés. Alors nous pourrions de dire que cet arc républicain suffirait à assurer le succès de cette proposition de loi, mais nous le savons jamais ne s'est jamais aussi simple que ça. Au Sénat, j'entends les réticences de Madame la rapporteure concernant la multiplication des délégations ou encore de groupes d'études, je suis d'ailleurs moi-même pour la rationalisation. Je les entends car là ce sont les mêmes depuis 20 ans. Les mêmes arguments qui en 2003 en 2009 en 2019 et maintenant en 2022, nous indiquait qu'il ne fallait surtout pas créer de nouvelles délégations et de nouveaux groupes d'étude. Et pourtant, chers collègues, je me suis penché sur les délégations que nous avons actuellement. Et si nous mettons de côté l'OPEX créée en 83 par la loi ou la délégation aux droits des femmes crient en 99 également par la loi. Nous avons depuis 2007 crée 5 délégations 2007 délégation renseignement 2009 délégations aux collectivités locales 2009 toujours délégation à la Prospective 2011 délégation aux outre-mer et la dernière et pas des moindres. 2014, création de la délégation aux entreprises créées par le bureau. Et donc en 20 ans, il n'est jamais le moment de créer une délégation aux droits de l'enfant et pourtant notre chambre a continué de créer légitimement un certain nombre de délégations utile au travail parlementaire. Mais la question de l'enfance, c'est pas une question annexe. L'enfonce par sa diversité par l'éventail des thématiques, elle regroupe est en soi un sujet majeur. Oui, chers collègues, les droits de l'enfant, ce n'est pas un sujet mineur.-- Sommes-nous capables de considérer les droits de l'enfant comme une priorité de nos politiques publiques et donc par définition un sujet transversal dans notre institution. Madame la rapporteure nous indiquera sans nul doute tous les travaux que notre chambre à mener sur le sujet de l'enfance et elle aura raison, nous avons beaucoup travaillé sur l'enfance. Mais je pense que si pourtant que nos travaux sur l'enfance ne doivent pas être une fonctionner en silos mais bien de façon transversale auprès des commissions permanentes. Il ne s'agit pas, comme certains le dénoncent d'une proposition et exclusivement symbolique bien sûr, il y a une dimension symbolique puisque la création d'une telle délégation aux droits de l'enfant enverrait un signal fort au monde de l'enfance qui demande cette création depuis plus de 20 ans d'ailleurs à l'inverse, un refus de la création de cette délégation enverrait un message catastrophique à l'opinion publique sur la chambre haute. Mais au-delà de cette portée symbolique. Il y a un enjeu beaucoup plus fort. Les délégations ont le temps de travailler sur le fond de prendre le temps d'alimenter par des auditions des rapports des travaux des parlementaires et des commissions pour mieux légiférer sur des rapports d'expertise. Par ailleurs, si nous passons la dimension symbolique qui est la dimension utile d'une telle délégation. Il faut rappeler qu'en ce qui concerne l'enfonce. Ce sont les départements qui sont chef de file, il s'agit donc d'une politique décentralisée. Il est donc souhaitable que le Sénat chambre des territoires et représentants des collectivités puissent s'intéresser sur ce sujet et son port fortement de cette politique. Je souhaiterais d'ailleurs prendre l'exemple de la délégation aux droits des femmes, qui effectue un travail remarquable, à l'image de son dernier rapport sur la pornographie. Cette délégation fonctionne bien par l'apport de ces réflexions de ces travaux et finalement alimente la réflexion du Parlement et de l'exécutif pour mieux légiférer. Il y a 33 ans, chers collègues. La France ratifie la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui nous obligeait à mettre l'intérêt supérieur de l'enfant au coeur de nos politiques publiques car chers collègues. Les enfants c'est pas seulement des petits être qu'il nous faut protéger les enfants, ce sont des sujets des droits à part entière. Alors cette depuis 1990, de nombreuses réformes législatives ont adopté en vue ont été adoptées en vue de mettre notre droit en conformité avec cette convention. Parmi les réformes figure notamment la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, celle de notre collègue Philippe Bas du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, celle de 2016 de Laurence Rossignol, s'appuyant sur les travaux de Michel Meunier ou encore la loi de 10 juillet 2019 relatives à l'interdiction des violences éducatives ordinaires et pour finir, celle portée par le gouvernement actuel en février 2022, beaucoup a été fait. Mais le constat reste alarmant, chers collègues. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, 25% des sans domicile fixe de moins de 25 ans ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. 70% des jeunes de la sortent sans diplôme. Les enfants sont les victimes directes ou indirectes des violences intrafamiliales ou encore de l'inceste qui démontre bien le lien entre la violence et la santé. 500 enfants de moins de six mois sont victimes chaque année du syndrome du bébé secoué qui par manque de prévention auprès des parents ou des tiers. Gardien 75 pour % des survivants ont des séquelles physiques ou mentales irréversible. 50.000 enfants sont victimes de violences physiques et psychologiques chaque année et près de 100.000 enfants ne sont pas scolarisés, 15 pour des jeunes en France connaissent un épisode dépressif caractérisé et ses amphis suicidaire qui malheureusement se concrétise parfois ont augmenté de 20% depuis la crise sanitaire. Le suicide d'ailleurs et la 2ème cause de mortalité entre les 10 25 ans.-- Sur les violences numérique. Ils sont souvent la proie d'agresseurs ultra-présent sur les réseaux sociaux avec la question sous fond du harcèlement. Je pense également aux problèmes de malnutrition au problème d'obésité 400.000 enfants porteurs de handicap sont scolarisés avec le défi de l'inclusion qui n'est jamais un long fleuve tranquille dans notre pays et qui malgré tout permet des vraies réussites mais aussi les inégalités sur le plan de la scolarité du sport et de la culture en particulier pour ceux qui sont en situation de handicap. Nous pouvons également parler des enlèvements parentaux à l'étranger et je sais que nous sommes nombreux sur cet dans cet hémicycle à être sollicités, interpellés par les parents victimes rester en France. Mais aussi le sujet des mineurs non accompagnés et l'impact que de cette augmentation sur ces dernières années sur. Nos départements et puis un chiffre. Enfin c'est glaçant. D'ailleurs mon signé par la commission des affaires sociales alors que son objectif davantage la commission des lois. Preuve de la transversalité ces sujets tous les 5 jours un enfant est tué. Par un de ses parents. Selon le dernier rapport de l'UNICEF. Mes chers collègues, tous ces sujets que je viens de citer, il en existe bien d'autres la question des droits de l'enfant est intrinsèque. Et pourtant ils sont traités indépendamment les uns des autres, dans les différentes commissions qui composent le Sénat. De non un cadre institutionnel aux parlementaires engagés sur cette cause comme je vous le disais, il s'agit d'un moment hein tordu. Important, attendu depuis 20 ans, attendu par les associations attendues par les parlementaires attendu par les professionnels, attendu par les enfants eux-mêmes et par l'opinion publique. Parce que la place de l'enfant doit être au coeur de notre société parce que le Sénat ne peut pas se détourner d'un travail de fond qui touchent directement nos territoires. Parce que je sais que nous avons tous envie de rentrer ce soir dans notre circonscription avec la satisfaction d'avoir été utile pour notre pays. Mes chers collègues, je connais tous votre engagement en faveur de la question des droits de l'enfant, que ce soit ici à Paris où chacun dans nos territoires en Europe pour l'international au sein de la Haute Assemblée comme à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi aujourd'hui, faisons ensemble le choix de nous tenir aux côtés de l'amélioration de la condition des enfants parce que les droits de l'enfant ne sont pas des droits mineurs chers collègues, je vous invite à soutenir la création de cette délégation aux droits de l'enfant. Je vous remercie. Merci cher collègue. Et la parole est maintenant à Madame, Muriel Jourda, rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes. Juin 2022 rapport d'information sur la lutte contre l'obésité. Octobre 2021. Audition de Monsieur Jean-Marc Sauvé, président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Octobre 2021. Proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie, nécessitent un accompagnement soutenu. Octobre 2021. Projet de loi relatif à la protection des enfants. Septembre 2021, audition de monsieur Adrien taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé chargé de l'enfance et des familles. Mai 2021 propositions de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. Décembre 2020, audition de monsieur Adrien Taquet. 5 février 2020. Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance au rayon audition de monsieur Adrien Taquet.-- Février 2022 rapport d'information établissant le bilan des mesures éducatives du quinquennat. Février 2022, proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire.-- Juin 2020, proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Juillet 2022, audition de Madame, Claire Hédon, février 2022 propositions de loi relative au choix du nom issu de la filiation. Janvier 2022, proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire. Octobre 2021, proposition de loi visant à réformer l'adoption. Mars 2021, audition de Madame, Claire Hédon.-- Janvier 2021 projets de loi ratifiant l'ordonnance du 11 septembre 2019, pourtant partie législative du code de justice pénale des mineurs. Janvier 2021, proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels et de l'inceste.-- juin 2020, audition de Monsieur Jacques Toubon. Défenseur des droits. Juin 2020, proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales. Avril 2020, audition de Monsieur Jacques Toubon. Janvier février 2020 cycle d'auditions sur le nouveau code de justice pénale des mineurs. Janvier 2022 propositions de loi vise à encourager l'usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d'accéder à Internet. Voilà pour les travaux des commissions des affaires sociales des lois et des affaires économiques. Travaux de la délégation aux droits des femmes. Septembre 2022 rapport d'information sur les industries de la pornographie. Juin 2022, table ronde sur la régulation de l'accès aux contenus pornographiques en ligne. Avril 2022 tables rondes sur la protection des mineurs face aux contenus pornographiques. Décembre 2021, audition de monsieur Adrien Taquet. Novembre 2021 tables rondes sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan. Novembre 2021, audition de Madame Catherine Champrenault de monsieur Charbonnier magistrats avril. Novembre 2020, audition de monsieur Adrien Taquet. Juillet 2020 rapport d'information sur le bilan de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au sein de la famille. Travaux communs des commissions permanentes, septembre 2022. Prévenir la déliquance des mineurs éviter la récidive. Septembre 2021 mineurs non accompagnés, jeunes en errance, février 2020 signalement par les professionnels astreint à un secret des violences commises sur les mineurs. Sur le président Madame la Ministre, mes chers collègues. Voilà une liste. Sans doute fastidieuse mais pas exhaustif des travaux que le Sénat, que les sénateurs ont mené depuis 3 ans, relatif à la situation des enfants. Pourquoi 3 ans parce que 3 ans c'est la date à laquelle notre collègue Madame la présidente, Éliane Assassi déposait une proposition de loi dans des termes similaires visant à créer une délégation aux droits des enfants. Cette proposition a été rejetée par. Le Sénat sur proposition de la commission des lois et j'étais d'ores et déjà rapporteur.-- Pourquoi cette énumération, vous l'avez sans doute compris compris aux propos de notre collègue Xavier il Iacovelli qui dépose à nouveau cette proposition de loi parce que la avis de la commission des lois a été à nouveau défavorable et je ne souhaiterais pas effectivement que cet avis défavorable soit interprétée comme un signal défavorable sur l'intérêt du Sénat face aux enfants. C'est pourquoi ce rappel du travail des sénateurs permet à mon sens 3 choses, d'abord de rappeler que nous travaillons souvent fréquemment sur la situation des enfants.-- De travailler que malgré l'absence de délégation. Nous travaillons aussi souvent de façon transversale et nous allons continuer à le faire puisque bientôt les délégations, droits des femmes et les délégations à l'Outre-mer va travailler sur la parentalité outre-mer. Et de rappeler que la création d'une délégation mais je ne pense pas que vous souteniez cela même si je n'adhère pas aux propos de Clémenceau qui dit que pour enterrer un problème, il faut créer une commission cette délégation ne résoudra aucun problème et nous le savons, ne serait-ce que parce que elle n'a pas comme les commissions législatives de pouvoir législatif. si cette proposition de loi et cette délégation n'a pas l'objet de faire travailler les sénateurs sur la situation des enfants puisque nous le faisons déjà si elle n'a pas pour objet de nous faire travailler de façon transversale puisque nous le faisons déjà, et si elle n'a pas de pour objet de résoudre une quelconque difficulté puisqu'elle ne possède pas de pouvoir législatif. À quoi sert cette proposition de loi, elle sert tout simplement à organiser différemment, a proposé une organisation différente du travail du Sénat. Je crois que nous l'avions déjà établi, lorsque nous avions étudié il y a 3 ans. La proposition de loi. La présidente, Éliane Assassi. Et personne ne s'y étaient trompés à commencer par la représentante du gouvernement à l'époque, qui avait indiqué clairement la décision de créer une délégation parlementaire est un sujet éminemment parlementaire, le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat et je vois mal quel autre position pourrait avoir d'ailleurs le gouvernement sur cette affaire. Donc nous sommes sur un sujet d'organisation de nos travaux. Là-dessus. Nous avons des précédents. Nous avons, je vous le rappelle, un rapport de 2015, rapport qui avait été établi par les présidents Roger Karoutchi et Alain Richard sur l'organisation de notre travail parlementaire et ce rapport avait conclu à quoi il avait conclu à l'arrêt de la police. c'est-à-dire de la multiplication des instances parlementaires qui apporte plus de dispersion que d'efficacité au travail sénatorial. Ce rapport, il avait été déposée. Devant le bureau du Sénat car en réalité l'organe l'organisation des travaux parlementaires, c'est le bureau et d'ailleurs la la l'Assemblée nationale qui vient de créer une délégation aux droits des enfants. La non pas on aime ici, comme nous sommes en train d'en discuter mais par une décision de la conférence des présidents qui est l'organe d'organisation de l'Assemblée nationale.-- Donc si nous souhaitons. Modifier cette jurisprudence qui est constante depuis 2015 et qui n'a pas été remises en cause par le bureau. Je vous invite ceux qui estimeraient nécessaire de créer cette délégation de vous en référer au bureau renverser cette jurisprudence de 2015 et cette position qui avait été unanime et qui n'a pas été modifiés depuis lors. Demander au bureau d'examiner cette création de délégation qui serait un nouvel organe de travail parlementaire permettrait je crois de remettre à sa place le débat car ne nous y trompons pas, nous parlons bien d'organisation de travail et nous ne parlons pas de la situation des enfants ni l'interdit de l'intérêt du Sénat portée à la situation des enfants car sur ce point l'intérêt du Sénat et je crois que l'énumération de nos travaux le démontre, a toujours été indéfectible. Je vous remercie. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur Xavier Iacovelli madame la rapporteure mesdames et messieurs les sénateurs. Avant toute chose, je tenais à remercier le sénateur Xavier il Iacovelli pour son engagement sans faille sur les sujets de l'enfance et je tiens aussi à remercier les signataires de cette proposition de loi qui nous permet une nouvelle fois et je m'en réjouis d'évoquer les droits des enfants, et plus largement la politique de l'enfance devant votre haute assemblée.-- Beaucoup a été fait au cours du précédent quinquennat avec en point d'orgue la loi du 7 février 2022 et je tiens ici à saluer le travail du Sénat. Notamment sur ce texte et tous les travaux que vous avez rappelé madame la rapporteure. Beaucoup a été fait mais il reste beaucoup à faire et les chiffres que vous avez rappelé monsieur le sénateur, rappelle une triste réalité, si on en retient quand un enfant meurt tous les jours dans le cadre familial sous les coups de vieux sous le coup, ce chiffre-là doit évidemment nous interpeller. Ils sont terribles. Ces chiffres et il nous rappelle que malgré les moyens humains et financiers engagés sur les politiques de l'enfance malgré les très nombreux acteurs engagés sur le terrain départements associations professionnelles de beaucoup de chant les droits fondamentaux de nos enfants sont encore fragiles, leur droit à la sécurité, leur droit à la santé. Leur droit au bien-être et au logement ou encore à l'éducation ne sont pas encore aujourd'hui assuré dans notre pays.-- Face à ce constat, nous devons inlassablement débattre, échanger réfléchir, agir. Et. Quelles que soient nos appartenances partisanes, quelles que soient nos champs de compétence. Pour chaque politique publique menée pour chaque texte voté nous femmes et hommes politiques adultes devons faire l'effort d'intégrer cette dimension, les droits de l'enfant de nos enfants sont-ils pris en compte. L'année prochaine. L'Organisation des Nations-Unies évaluera la France au regard des exigences de la convention internationale des droits de l'enfant. Nous devons nous devrons être à la hauteur. Le pays de droits de l'homme, le pays des droits de la femme doit démontrer qu'il est aussi le pays des droits de l'enfant.-- La mobilisation de tous. C'est donc une nécessité je dirais aujourd'hui une urgence. Vous le savez l'engagement du gouvernement est très fort. Le président de la République a souhaité faire de l'enfance et de sa protection. Un des sujets prioritaires de ce quinquennat.-- Cette priorité a été au coeur du 1er comité interministériel de l'enfance au lendemain de la journée internationale des droits de l'enfant.-- Avec la Première ministre les nombreux ministres concernés ont déterminé 5 chantiers prioritaires et une quarantaine de mesures dont il m'appartiendra de coordonner la mise en oeuvre.-- Je tiens ici à vous en présenter quelques-unes. La première des priorités, c'est bien sûr la lutte contre les violences faites aux enfants. Dès l'année prochaine. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin créera un office de police judiciaire spécialisés. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti publiera une circulaire de politique pénale accompagnons cette création.-- Le second chanter c'est celui de la santé en ce compris la santé mentale de nos enfants. C'est un sujet prioritaire et vous le savez sur le terrain, c'est un sujet de grande préoccupation, qui remonte à chacun de mes échanges notamment avec les présidents des départements.-- Le ministre de la Santé François Braun a lancé hier les assises de la santé des enfants et de la pédiatrie qui permettront au printemps de définir des orientations très attendu.-- 3ème priorité le numérique partout où sont nos enfants, nous devons les protéger et notamment sur Internet. C'est pourquoi la loi Studer sous le contrôle parental sera effective dans les prochaines semaines nous lancerons à cette occasion avec Jean-Noël Barrot, une campagne de communication pour accompagner les parents dans cette parentalité numérique si complexe.-- Mais au-delà de l'engagement de tous les ministres, je sais que vous serez sensible mesdames et messieurs les sénateurs. Il nous faut renforcer notre action aux côtés des départements pour que les enfants les plus fragiles, notamment les enfants en situation de handicap ou ceux de la protection de l'enfance est un accès facilité à tous les dispositifs de droit commun. L'État doit être en effet plus fort aux côtés des départements et des acteurs de terrain.-- Il doit être présent en les accompagnant, financièrement, contractuels. Contractualisation mais aussi en renforçant avec les préfets, la coordination de l'ensemble des administrations et des services de l'État sur les sujets de l'enfance.-- La loi du du 7 février 2022 a donné la possibilité d'expérimenter des comités départementaux de protection de l'enfance qui sous l'égide du préfet et du président du département peut réunir l'ensemble des acteurs engagés.-- Les fameuses direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité. L'éducation nationale, la santé, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse en présence de l'autorité judiciaire.-- Je crois beaucoup à la mise en place de ces comités départementaux qui correspondent à un vrai besoin de terrain pour améliorer la stratégie de l'offre. Les contrôles et évidemment derrière tout ça, la qualité des parcours des enfants notamment ceux en situation complexe.-- Et ce constat est largement confirmé par mes échanges avec les élus et les acteurs locaux je tiens donc à débuter cette expérimentation dès janvier prochain. Je souhaite maintenant souligner combien les parlementaires sont aussi très engagé sur les sujets de l'enfance. Ce débat, on est une manifestation évidente, je l'ai dit.-- Depuis ma prise de fonction, il y a six mois, je l'ai con je le constate lors des travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale récemment lors de l'examen du projet de loi de finances mais également lors des rendez-vous que j'ai avec vous et ils sont nombreux et à l'occasion de mes déplacements sur le terrain.-- L'Assemblée nationale a fait le choix de créer en septembre une délégation parlementaire aux droits de l'enfant.-- Comme vous le savez j'ai salué la création de cette délégation.-- Si aucun ministre n'a le monopole de l'enfance. Moi non plus. Il en est de même pour les travaux des assemblées et de leur commission. Le sujet de l'enfance peut en effet et être être abordée dans plusieurs commissions. Je dirais même il doit être abordée dans plusieurs commissions celle des affaires sociales naturellement mais aussi celle de la commission des lois, ou encore la commission des affaires culturelles et de l'éducation.-- Les droits de l'enfant sont partout, mener la transition énergétique n'est-ce pas avant tout préparer l'avenir de nos enfants. Ce sujet faire des droits de l'enfant. L'affaire de tous, mettre toutes les politiques à hauteur de nos enfants me tient pleinement à coeur et je veille tant au sein du gouvernement que sur le terrain à favoriser les échanges entre les acteurs dans un souci permanent de partage de l'information et d'efficacité.-- Au sein du Sénat la délégation aux droits des femmes, donc je salue la présidente et les membres je vous par exemple un rôle précieux en ce sens les travaux récents sur la pornographie ont fortement démontrer et je m'a pu régulièrement dessus.-- Toutefois, je l'ai d'ailleurs dit aussi à l'Assemblée nationale et je le répète, au Sénat, une création de délégation relève de l'organisation interne des travaux du Parlement. Je ne peux que m'en remettre à la sagesse de votre outre assemblée. Je voudrais renouveler ici ma volonté de travailler avec vous toutes et tous et ce quelle que soit la décision que vous prendrez à l'issue de l'examen de ce texte. Je sais que chacune de vos commissions quel que soit votre vote seront attentives seront encore plus attentive à intégrer les droits des enfants à leurs travaux.-- Car je le sais. Nous sommes toutes et tous pleinement engagés et s'il y a bien un sujet qui doit nous rassembler, c'est celui de l'avenir de nos enfants, je vous remercie. À la suite de la discussion générale. La parole est d'abord à madame Mélanie Vogel, pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour 4 minutes. Si. Monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues, bon la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui est assez simple, il y a un nombre conséquent de sénateurs et de sénatrice de tous les groupes ou presque qui souhaiteraient comme les députés travailler sur la question des droits de l'enfant au sein d'une délégation dédiée. Est ce qu'on pense que c'est utile, auquel cas on vote pour cette proposition de loi ou est-ce qu'on pense que ça ne sert à rien et auquel cas on vote contre. Donc. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je crois que c'est utile et pourquoi les écologistes voteront évidemment ce texte. La demande de création d'une délégation sénatoriale aux droits de l'enfant, c'est une demande de longue date des associations qui dans ce pays travaillent sur la question de l'enfance et qui est soutenu de manière transpartisane au Sénat. Pourquoi. Bah, d'abord parce que la situation des droits de l'enfant en France. c'est pas glorieux inceste. Pédocriminalité violence santé physique et mentale pauvreté alimentation sport handicapées inclusion éducation questions pénales il y a tellement de sujets qui doivent être regardée. Du point de vue spécifiques des enfants. Je voudrais prendre un exemple. Celui de l'inceste. Il y a 160.000 victimes d'inceste par an ça en moyenne 2 enfants par classe. C'est un phénomène massif auquel à ce jour aucune politique publique n'a su répondre. Je crois qu'il faut regarder les choses en face, on ne sait pas gérer, on ne sait pas faire le nombres d'inceste en France ne diminue pas et on ne sait pas faire en partie parce qu'on ne part jamais du point de vue des enfants victimes. On dit par exemple qu'il faut que les enfants parlent mais on ne prend pas en compte le contexte qui fait que les enfants ne parlent pas le système qui est l'inceste c'est logique propre les logiques de son omerta sociale ni les impacts que vont avoir le fait de parler pour les enfants ou les adultes qui le font. Puis on insiste sur la réponse pénale, le problème c'est terrible on aimerait tellement que ce soit si simple c'est que la perspective de la prison n'empêche pas les insectes et la prison n'empêche pas les récidives aussi sans partir du point de vue des enfants concernés. On construit des politiques publiques qui gère l'existant. Des victimes brisé et des violeurs on fait parler les enfants et on emprisonne parfois les autres mais on ne fait pas baisser le nombre d'inceste en France et je crois qu'on pourra jamais construire de politiques publiques satisfaisante sans avoir mené un travail en partant du point de vue des enfants lorsque ça les concerne. Et c'est ce qu'une délégation permis la création d'une délégation parlementaire dédiée à un sujet permet de se concentrer sur un point de vue qui sinon est noyé et au fond jamais pris en compte. Ça permet de creuser des sujets spécifiques via un travail d'information, d'enquêtes de recherche au-delà du travail législatif et c'est ce que les délégations qui travaillent montrent tous les jours. Toutes les raisons semblent donc réunis pour être favorable à cette loi, pourtant la commission des lois, s'y oppose au motif par exemple que le sujet déjà traité ailleurs notamment par la délégation aux droits des femmes. c'est un problème parce que il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne sont pas de futur femme il y a pas que des femmes qui ont des enfants, donc on s'accordera sur le fait qu'il a pas nécessairement un grand lien. Par ailleurs, bien sûr il y a toujours un travail de commission sur les sujets de l'enfance Affaires sociales loi culture éducation et ça continuera mais éparpillés ici et là nous perdons l'intérêt politique de créer un espace espace de travail qui prennent comme perspective première l'intérêt de l'enfant et qui réfléchissent aux différentes politiques publiques de ce point de vue. Le 2ème argument c'est qu'il ne faut pas multiplier les délégations. D'accord. Mais enfin on a créé en 2014 au Sénat. Une délégation aux entreprises. Alors c'est très bien, j'ai rien contre la délégation aux entreprises. Je suis sûre qu'elle fait un très grand travail mais est-ce qu'on est en train de dire que les entreprises ont un besoin transversale d'être étudiés en dehors des commissions des sénats sous peine d'être l'angle mort des politiques publiques et que les enfants non franchement je crois pas que ce soit très sérieux. aujourd'hui que nos collègues. Merci à l'Assemblée nationale se sont dotés d'une délégation aux droits de l'enfant. Je crois que montrer aujourd'hui notre soutien à cette loi participerait à montrer que le Sénat n'a pas une volonté perpétuel de s'opposer à toutes les avancées sociales. Je vous remercie.

Monsieur le président, madame la ministre madame la rapporteure, mes chers collègues. La proposition de loi de notre collègue Xavier Iacovelli propose d'inscrire dans la loi la création de délégation parlementaire aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle fait le constat largement partagé sur nos bancs comme dans la société civile que de nombreux défis restent à relever pour assurer le respect des droits de l'enfant dans notre pays. Ce n'est pas la première fois que des initiatives législatives sont prises en ce sens en 2003 à l'Assemblée nationale se saisissait déjà de cette question en adoptant sans toutefois qu'elle ne prospère, une proposition de loi de Jacques Barrot et de Dominique Paillé. Plus récemment, en 2019, d'une proposition de loi du groupe CRCE était rejetée par le Sénat qui, suivant l'avis de la commission des Lois avait estimé que notre chambre se saisissait déjà pleinement de ces sujets et était en mesure de veiller efficacement au respect des droits de l'enfant. la position de la commission n'a pas changé depuis. Comme en atteste l'avis défavorable de la rapporteure. Le contexte politique, lui, n'est plus tout à fait le même. Je ne reviendrai pas sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement et encore tout récemment par la Première ministre, vous le savez madame la ministre. Et vous l'avez rappelé quelques instants je rappellerai seulement. En faisant mien l'un des constats d'UNICEF France. La persistance d'inégalités tant sociales que territoriales en particulier dans les quartiers prioritaires de la ville et les territoires d'outre-mer qui empêche un trop grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'école au service de santé ou de protection. Vous savez mon attachement à ce sujet. Les arguments qui te plaît d'en faveur de la création de délégation parlementaire aux droits de l'enfant sont nombreux. Une délégation un cadre à des travaux approfondis et transversaux sur des questions jusqu'à l'heure inexplorée ou abordé de façon parcellaire. Je pense notamment à la santé mentale des enfants ou à la pauvreté infantile sur lesquels il nous faut avancer. Une délégation. C'est aussi une visibilité supplémentaire offerte aux travaux du Sénat. L'écho médiatique dont ont récemment bénéficié les rapports de la délégation aux droits des femmes et là pour le prouver, la création d'une délégation aux droits de l'enfant au Sénat faciliterait par ailleurs les échanges avec l'Assemblée nationale et le Parlement européen et permettrait un meilleur suivi Et l'alimenterait enfin dans le respect bien sûr de la séparation des pouvoirs, la réflexion du gouvernement, en vue notamment de l'envoi du rapport périodique de la France au comité des droits de l'enfant des États Unis Ce sont ces arguments et ceux avancés tout à l'heure par notre collègue Xavier Iacovelli qui ont présidé à la création, en septembre dernier d'une délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée Nationale ce texte propose. Au Sénat, de limiter en inscrivant dans la loi. Cette initiative parlementaire. Le groupe RDPI votera naturellement en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est maintenant à la présidence, Laurence Rossignol, pour le groupe socialiste écologiste. Et républicain et pour six minutes. Madame la ministre madame la rapporteure, chers collègues, je vais vous lire un petit extrait dont je vous dirais ensuite de quoi il est issu. L'article 43 de la Constitution établie au demeurant la compétence des commissions pour l'examen des projets et propositions de loi. Cependant, la fragmentation des compétences illustrent le caractère transversal de la question de l'égalité des droits. Elle peut entraîner un défaut préjudiciable à une vision globale et constituait un obstacle. L'examen de textes successifs par différentes commissions peut ne pas pleinement permettre d'intégrer l'objectif d'égalité entre les sexes Bon je comprends que ça vous donne, je n'arrive pas à capter votre attention. Ce que je voulais vous dire c'était le rapport de la commission des lois en 1999 lors de l'adoption de la proposition de loi et non pas d'une décision du bureau de la création de la délégation aux droits des femmes. il semblerait que parfois la commission des lois varices. Vous avez Madame la rapporteure égrainé les différents travaux du Sénat travaux législatifs qui ont concerné des enfants. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez démontrer en réalité. Que le sénat examine les propositions droit et les projets de loi concernant les enfants bon côté, c'est bien le moins quand ils arrivent sur son bureau. Que le Sénat, parfois même. Propose des évolutions législatives c'est bien le moins encore c'est notre travail. Et puis enfin vous avez cité abondamment les rapports de la délégation aux droits des femmes. J'en espérais pas tant. Justement la délégation aux droits des femmes à laquelle je participe depuis que je suis sénatrice aimerait bien ne plus être chargé de s'occuper aussi de la question des enfants. Voyez-vous le sens même de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'émancipation des femmes consiste aussi à nous émanciper de la charge mentale des enfants y compris en délégation. Donc nous ne voulons plus de ça. Il y a exactement 98 ans, la société des nations adoptait la déclaration de Genève sur les droits de l'enfant. J'imagine que si c'est de leurs auteurs assistaient à nos travaux aujourd'hui à notre débat il serait stupéfait. D'observer qu'une délégation aux droits de l'enfant au Sénat en 2022 rencontrent toujours autant d'opposition d'incompréhension et j'ai presque envie de vous dire d'ignorance. Parce que je crois que votre propos qui n'est pas un propos sur la forme, je suis. Pas une petite poulette de l'année et il y a longtemps que j'ai compris que les débats de forme car j'en réalité des oppositions de fond la question n'est pas celle de nos travaux notre surcharge ou de l'organisation. Mais est-ce que vous êtes ou non d'accord pour que les droits de l'enfant soit un sujet traité de manière permanente par notre assemblée. Et je crois que vous ne savez pas ce que c'est que les droits de l'enfant a été les droits de l'enfant. Ce sont d'abord ses besoins. Ses besoins dans leur approche multidimensionnelle. Les besoins de l'enfant et les politiques publiques qui vont garantir son bon développement tant sur le plan social qu'individuelles tout en lui permettant de vivre pleinement ce temps privilégié qu'est le temps de l'enfance. Et crée une délégation aux droits des femmes, c'est affirmer la cohérence d'une stratégie globale pour l'enfance une stratégie décloisonner. Et dont l'objectif est de mettre en oeuvre des politiques publiques favorables au développement de l'enfant dans ces 5 dimensions.-- Qui sont physique affectif, intellectuel moteur et sociale et dans le respect de ses droits également les droits de l'enfant des écoute de ces besoins fondamentaux des enfants crée une délégation aux droits de l'enfant ici au Sénat c'est nous doter d'une capacité d'expertise pour agir au plus près des réalités présentes des enfants et de leurs familles et c'est anticiper pour s'adapter les transformations familial alors je sais que les transformations familial ont un peu tendance à électriser cette assemblée et à créer des réactions un peu tendu. Pour autant, elles existent et ce n'est pas ici qu'on décide. Transformation familial ici on ne fait que les accompagner et garantir que les transformations familial respecte l'égalité des membres des familles et les droits de l'enfant, c'est ça notre travail, ce n'est pas les deux les transformations sociétales des transformations économiques, elles sont à l'oeuvre. Et aussi créé une délégation à de l'enfance et permettent de décloisonner des politiques publiques aujourd'hui l'enfant la politique de l'enfant sont sectionnés. Vous avez l'éducation vous avez politique familiale, vous avez le sport, vous avez la santé. Or les besoins des des droits de l'enfant nécessite une approche panoramique en appui justement sur son développement multidimensionnel. Un enfant c'est la combinaison de différentes sphères de vie. Je sais que là encore, je vais choquer. On aimerait tellement que l'enfant ne soit que l'objet de sa famille que seule la famille et des parents puissent avoir la main sur le développement d'un enfant mais ce n'est pas le cas, un enfant il est la combinaison de ces relations aux parents de la vie à la maison de la vie dans la ville dans la nature, les loisirs, le sport, la culture, sa citoyenneté, aussi on en parle. Sa protection contre les violences sexistes et sexuelles. Écran contre la pauvreté. C'est tout ça la politique des droits de l'enfant et c'est tout cela que nous voulons-nous sénatrice des sénateurs moderne.-- Accompagnant un mouvement commencé il y a 100 ans à la société des nations.-- Traité au Sénat nous voulons pouvoir apporter notre capacité sertis. Nous sommes le chaînon manquant entre les associations et les politiques publiques. Il manque le Parlement. C'est la première fois que je vous entends, chers collègues. Dire qu'en fin de compte, le Parlement doit se dessaisir d'un sujet ou d'une compétence en la laissant soit la société civile soit au gouvernement. Non, non, nous voulons une délégation droits de l'enfant.

Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, l'enfant a le droit au respect de sa dignité et de son amour propre au respect pour chaque minute qui passe, comme l'écrivait le célèbre au pédiatre polonais Janusz Korczak inspirateur et précurseur de la convention des droits de l'enfant. Le groupe CRCE et par son engagement constant en faveur des droits de l'enfant s'inscrit dans une telle conception. Rappelons qu'en France et par la loi du 9 avril 1996 que le Parlement français décide de faire du 20 novembre. La journée nationale des droits de l'enfant initiative issue d'une proposition de loi des sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, adoptée le 14 octobre 95 à l'unanimité. Aussi, nous soutenons la proposition de loi initiée par notre collègue Xavier Iacovelli visant à créer une délégation parlementaire aux droits de l'enfant en souhaitant très franchement, mes chers collègues, qu'elles ne subissent pas le même sort que si identique dans notre groupe projeté le 20 novembre 2019, ici même. Alors pourquoi examiner à nouveau une telle PPL tout simplement parce que 33 ans après l'adoption de la convention internationale des droits de l'enfant. Ceux-ci ne sont pas toujours respectées en France dans notre pays, un enfant sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté, soit près de 3 millions d'enfants en 20 ans le nombre d'enfants de moins de 18 ans ans vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 16 à 20%. Ainsi des dizaines de milliers d'entre eux vivent et dorment dans la rue. Nous ne pouvons ignorer non plus les inégalités en matière de santé, de logement, d'accès à l'éducation ou aux loisirs qui demeure extrêmement Je ne peux ici qu'exprimer mon à mon inquiétude et celle de mon groupe concernant des enfants étrangers nés en France où se arrivés seuls ou avec leurs parents qui vivent des situations particulièrement difficiles contraint à une vie précaire placé en centre de détention de rétention expulsés avec leurs parents. Je tiens d'ailleurs à dénoncer le manque d'action de l'État face aux mineurs installés dans un campement à Ivry et depuis quelques jours devant le Conseil d'État. Le fait qu'ils soient étrangers ne peut en aucune façon expliquer ou pire. Cette situation intolérable est profondément inhumaine. Nous ne sommes pas dans la France de Zola mais au 21ième siècles, mes chers collègues. Réveillons-nous c'est inhumain. Et puis en matière de justice, on assiste à un durcissement pénal depuis le nouveau code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, qui remet profondément en cause l'ordonnance de 1945 et la primauté des mesures et éducatives. Un enfant est un enfant. Pour toutes ces raisons, nous devons agir. Le Parlement doit être à l'initiative d'une veille et d'un contrôle plus assidus du respect des droits des enfants. À l'heure des scandales qui éclatent sur les violences. Les agressions sexuelles des incestes nous devons ici au Sénat, a montré une détermination sans faille afin de créer les conditions d'un travail rigoureux sur les droits des enfants. C'est ce qu'ont fait fort à propos. Nos collègues de l'Assemblée nationale le 13 septembre 2022 examiner des propositions de loi des projets de loi, avec le travail spécifique d'une délégation ne peut être qu'un plus, je le vois parfaitement, ça a été dit-il dans la délégation aux droits des femmes qui n'empiètent aucunement sur le travail des commissions qui sont saisis au fond tout en apportant une plus-Value et une expertise. Et puis le propre d'une délégation, c'est précisément de traiter des sujets transversaux. Je ne partage donc pas madame la rapporteure. Vos arguments sur la rationalisation des structures ou le renvoi de la décision au bureau du Sénat c'est fuir ses responsabilités, c'est donner une image rétrograde du Sénat. La France pays des droits de l'homme doit se montrer sur ce point exemplaire dans l'effectivité des droits de l'enfant et leur enrichissement la protection de l'enfance est un sujet primordial que nous partageons ici sur le banc et avec Madame la Ministre une délégation droits de l'enfant serait un signal fort envoyé aux associations, aux enfants de la zone à tous les actes à toutes les actrices et les acteurs impliqués sur cette question et qui veulent être entendus. Nous voterons donc cette PPL et j'espère que nos collègues hésitants vont nous suivre. Merci cher collègue. Il est à présent monsieur Philippe. Bonnecarrere pour le groupe Union centriste et pour six minutes. monsieur le Président Madame la Ministre de même rapporteur chers collègues après un certain nombre de présentation passionnée et. Ou enflammer. Nous voyons bien que nous sommes en train de reconstituer les les débats de de notre enfance ou les rédactions de notre jeunesse sur le thème du coeur et de la raison.

Les voix de la raison. Se rend moins apprécié que les voix du coeur parce que au bout du bout, qu'elle est effectivement le le Est-ce que il y a un débat au regard de l'intention de chacune et chacun d'entre nous. À l'égard des droits de l'enfant ça autorisé moi vous le contestez totalement pour moi il n'y a aucun débat de près ou de loin sur l'un ou l'autre des bancs les bancs du. Sénat, la préoccupation est la même, il n'y a pas pour dire plus franchement des choses de débat entre des conservateurs ou des modernistes sur la question des droits de l'enfant. Il y a.-- À cet égard. Illimité. Reste la question qui est quand même celle qui est au coeur de toute action publique, de savoir comment. On traite les sujets et comme on essaie d'avoir l'accent de public la plus efficace, il y a 2 options en ce qui concerne en tout cas les travaux parlementaires, l'une qui consiste à flécher une délégation suisse Icic. Au delà des groupes d'études éventuelle l'autre qui considère que l'Organisation parlementaire par ce structure par les commissions. Qui sont susceptibles de traiter des sujets a déjà sonne son efficacité, les 2 arguments peuvent effectivement se valoir. Pour prendre un mot qui a été utilisé par. Madame Bougel qui était le mot éparpillement j'aurais failli utiliser le le le mot émiettement elle nous a dit. N'éparpillés pas le sujet entre les différents sur deux entre les différentes commissions. Vous voyez bien que vous avez besoin d'une délégation pour éviter cet effet d'éparpillement envers de cette situation si vous créez sur chaque sujet transversal. Une délégation. Alors vous êtes bien dans l'éparpillement ou de l'émiettement puisque vous aimiez étiez l'action parlementaire entre différentes structures et vous savez également, il n'est pas interdit de se dire les choses. En toute réalité de vérité chers collègues que entre les débats dans. L'hémicycle. En séance, le suivi des commissions. Le suivi des délégations. Vous êtes amené les uns et les autres à courir après votre agenda, il y a aussi des limites de cette à l'exercice. je ne suis pas certain que la multiplication des délégations souhaitent une réponse et plus particulièrement, j'aurais tendance à me méfier la soeur j'assume complètement. C'est cette responsabilité je méfie de tout ce qui concerne les notions d'affichage. madame Cohen a terminé son propos en indiquant qu'il fallait envoyer des signaux. Cette idée que la vie publique passerait par le fait d'envoyer des signaux passerait par les journées mondiales de ceci ou de cela, est une idée que je ne crois pas pertinente. Ça c'est des logiques d'émotion, ce sont des logiques de de de communication c'est un peu parallèle et il y a pas de hasard, au fait que cette question était un moment évoquée dans les présentes interventions. À la question de l'inscription. De toutes les normes juridiques dans notre dans notre Constitution. À quel moment on est dans l'action publique. À quel moment on est dans l'affichage. Il me semble qu'il peut y avoir un abus des dispositions d'émotion ou des dispositions. Et c'est ce qui fait que, majoritairement de notre groupe, même si je ne vous cacherai pas parmi nos collègues un certains nombres soutiennent effectivement cette idée de la délégation aux droits de l'enfant et l'ont portée depuis depuis le début. Donc, il ne semble pas ma chère collègue que des propos comme qui. Ce sont ceux de la même le rapporteur ou de votre serviteur demandant simplement ce qu'on puisse travailler de la manière la plus raisonnables plus efficace dans notre dans notre doit poser difficulté dans les arguments s'il m'est possible. De faire sourire éventuellement d'notre président de séance qui ont je regarder le rapport rédigé par la même Jourdain je voyais qu'il était fait référence à un rapport du Bureau sur les méthodes de travail du du Sénat qui nous avait invités à éviter la dispersion des sénateurs

ce lexique. Soit suffisant à répondre aux préoccupations mais plus sérieusement. Pour revenir à la question évoquée notre assemblée mène de nombreux travaux je ne comprends pas ce qui a été ce qui a été évoqué tout à l'heure par plusieurs intervenants. Donc il y a un contrôle soutenu sur les sujets les plus variés. je ne veux pas rajouter encore des arguments mais quand j'entendais puisque j'écoute les collègues mais c'était au Chili. Il y a quelques minutes. Indiqué qu'il fallait avoir un meilleur suivi de l'application des lois dans le domaine des droits des enfants. Et vous savez bien que c'est une question qui est posée à l'ensemble de notre assemblée que celui de la meilleure le meilleur suivi des lois. Cela vaut pour la question des droits des enfants. Comme pour tous les autres sujets, donc je ne pense pas que notre assemblée est à rougir du. De son travail continue la multiplicité des travaux réalisés le démonte. Je ne pense pas qu'elle ait à rougir de sa capacité. À assurer la transversalité au bout du bout, chacun prendra bien sûr ses responsabilités Madame Rossignol par. Ah pardon, effectivement je l'avais pas vu que je dépassé le temps de parole, je vous prie d'un accusé, votre observation est parfaitement justifiée. Merci. Merci cher collègue. Madame Benbassa la parole pour le groupe des sénateurs. Enfin pour les sénateurs. N'appartenant à aucun groupe. Et à la trois minutes.-- Monsieur le Président Madame la ministre. Madame la rapporteure, mes chers collègues, la création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant se heurte. Une nouvelle fois au refus d'un grand nombre de nos collègues de la commission des lois. Les raisons que celles-ci évoque, vous m'excuserai sont peu argumentée. Comme en 2019 vous justifier le rejet de ce texte par des considérations relatives à la méthode du travail parlementaire. Nous avons été élus pour porter la voix de nos concitoyennes concitoyens et de nos collectivités. Les services de l'aide sociale à l'enfance sont saturés et manquent de moyens pour agir. Par exemple, en novembre 2021 un nourrisson âgé de seulement 13 mois est décédé. Battu à mort par ses parents, alors même qu'il faisait l'objet d'un signalement et qu'il bénéficiait d'une mesure de protection de l'enfance. Ce drame aurait pu être évité. Je pourrais vous citer tellement de tragédies liées à l'inceste et à la maltraitance qui se finissent ou par un suicide ou par un coup mortel en l'occurrence la responsabilité de l'État est immense. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales met en évidence un enchaînement de circonstances défavorables et de défaillance profonde dans le système de l'ASE. En plus de son dernier rapport accablant la défenseure des droits Claire, Claire Hédon s'est saisi le 15 novembre dernier de la situation alarmante et préoccupante des mineurs placés dans le nord et et la somme les juges des enfants de ces départements ont alerté sur le manque de places en foyer sur des placements non exécuté des mesures d'assistance éducative non pris en charge avec des délais excédant les six mois. Ainsi une véritable rupture s'opère entre les enfants laissés pour compte et l'État largement désengagé la défenseure des droits l'affirme la protection de l'enfance n'est plus dûment. Dans certains territoires selon la, la Fondation Abbé Pierre. Un quart des personnes SDF aujourd'hui sont d'anciens enfants placés. Vous voudriez alors nous faire croire qu'il n'est ni légitime, ni efficace ni cohérent de créer cette délégation parlementaire aux droits de l'enfant, que ça soit dans les domaines de l'éducation de la santé, notamment depuis l'épisode de Covid de la justice et aussi de la protection de l'environnement. Les enfants ont une place à part entière dans nos politiques publiques. Engageons-nous réellement dans cette cause et Cléon enfin cette délégation qui serait une fenêtre ouvert du Parlement pour y faire entrer la enfant à part entière un organe d'action. Et de proposition, je voterai ce texte et je remercie. Le. L'auteur de la PPL, monsieur Iacovelli. Donc, la parole est à madame Maryse Carrère pour le groupe. Du Rassemblement démocratique social et européen.-- Monsieur le président, madame la ministre madame la rapporteure monsieur l'auteur de la proposition de loi, mes chers collègues. Il y a quelques jours lors de l'examen du budget, j'avais l'occasion de dire certaines difficultés auxquelles étaient confrontés les services qui gravitent autour de l'accompagnement de la enceinte. Entre surcharge de travail, manque de moyens et de personnel et un engagement de plus en plus conséquent face aux situations de plus en plus complexe et douloureuse. La protection de l'enfance de main-d'autant de persévérance que de patience et j'en profite pour rendre hommage à ceux qui s'y dévouent souvent pour des salaires modestes et des emplois du temps Je voudrais remercier Xavier Iacovelli de son initiative. Elle doit nous maintenir un alerte. On pourrait considérer que sur la forme, cette proposition de loi pose une difficulté d'autant que notre groupe n'est pas toujours favorable à l'inflation législative. Certes l'objectif poursuivi par ce texte pourrait être atteint autrement que par une loi comme ça a été le cas à l'Assemblée nationale. Notre conférence des présidents pourrait se charger elles-mêmes de la création d'une délégation aux droits des enfants. Mais à défaut. Il fallait trouver un moyen de l'alerter. Cette proposition de loi le permet. S'agissant du fond maintenant. Il est légitime de s'interroger sur la nécessité d'une telle délégation qui dans cette Essimi dans cet hémicycle n'est pas favorable à ce que nous portions une attention, une attention particulière à la question des droits de l'enfant évidemment personne est loin de nous l'idée de renier tout le travail réalisé ces dernières années. Il va de soi que la demi-de que la définition de l'intérêt de l'ensemble peut varier de pris à l'autre mais sur les sujets les plus fondamentaux, nous savons être unanimes. Je pense par exemple au texte qui avait porté notre collègue Annick Billon, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste et et chacun se souvient d'ailleurs de l'injuste traitement médiatique dont elle avait été l'objet.-- Il est clair qu'aujourd'hui notre hémicycle apporter à ce moment-là une avancée significative dans la lutte contre et violences sexuelles faites aux enfants, même si il reste des progrès encore à faire aussi pour revenir au texte du jour notre rapporteur l'a souligné le Sénat défend déjà et depuis longtemps les droits et l'intégrité des enfants nos nombreux travaux en témoigne notre rapporteur a pu refaire la liste non exhaustive des rapports et auditions de ces dernières années, ça ne fait l'objet d'aucun débat. C'est un sujet sur lequel nous travaillons. Toutefois, malgré ces éléments, je n'irai pas dans le sens de notre commission d'ailleurs quelques membres du groupe RDSE ont aussi co-signé cette proposition de loi au contraire puisque c'est un sujet majeur. Plutôt que de multiplier les initiatives et plutôt que d'éparpiller nos réflexions. Pourquoi ne pas structurer cet ensemble au sein d'une même structure cette délégation droits des enfants. Personne ici ne dira que les autres délégations déjà institué manque d'utilité et de légitimité, elles permettent d'offrir des réponses et des analyses transversales marquée par la spécialité et l'expertise sur une thématique qu'il s'agisse de la décentralisation de l'égalité des chances des entreprises ou encore de l'outre-mer. Elles sont aussi des lieux de dialogue et d'analyse prospective de grande qualité qui viennent nourrir nos travaux législatifs. Alors pourquoi pas une délégation aux droits des enfants. Je n'ai aucun doute que cette nouvelle délégation trouverez toute sa place dans notre hémicycle aussi notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi. Monsieur le Président Madame la Ministre. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. À l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant le 20 novembre dernier, l'UNICEF a publié des chiffres alarmants. En France, un enfant est tué par l'un de ses parents, tous les 5 jours en moyenne et l'association enfant Bleu a pour sa part constaté une augmentation de 45% des appels de victimes ou pour témoigner de maltraitance sur des enfants en 2022 par rapport à 2029. Ainsi forcé de constater que si la France progresse en matière de protection des enfants. Elle n'a pas encore réussi à éradiquer les violences faites à leur encontre et à faire respecter leurs droits. Quelque 3 millions d'enfants vivent en France sous le seuil de la pauvreté et les inégalités en matière de santé, de logement, d'accès à l'éducation ou aux loisirs demeure bien trop conséquente. S'ajoute à cela de nouvelles formes de violence physique mais aussi morales tels que de harcèlement la maltraitance la pédophilie l'exploitation sexuelle dans le cadre familial. Bien souvent, mais aussi et de plus en plus dans le cadre scolaire et ou médico-social. La situation est bien plus dramatique dans le monde. La guerre, la misère et la pauvreté, les inégalités et le changement climatique mettent en péril la vie de millions d'enfants. Ayant mes chers collègues, en tête ces données très préoccupante alors que nous examinons aujourd'hui la proposition de loi tendant à la création de délégation parlementaire aux droits de l'enfant. Plusieurs collègues ont ici rappeler c'est la convention internationale des droits de l'enfant adopté par les Nations-Unies. Le 20 novembre 89 et que la France a ratifié en août 1990, qui garantit les droits interdépendants et inaliénable des enfants. Le texte vise la protection spécifique de l'enfant en tant que sujet de droit à part entière sont ainsi pris en considération le caractère vulnérable et la nécessité de développement de l'enfant. Il a ainsi droit à une identité droit à la santé à l'éducation à une vie de famille à un niveau de vie suffisant droit d'être protégé de la violence. Droit de s'exprimer. Droit d'être protégé de la guerre d'être protégé de l'exploitation droit de jouer. Droit d'avoir des loisirs. Trois protocole facultatif ont complété cet instrument entré en vigueur en 2014 et 2022. Ils concernent notamment l'implication des enfants dans les conflits armés et la nécessité de les protéger contre leur recrutement, ils entendent également lutter contre la vente d'enfants la prostitution, la pornographie, les mettant en scène. Pour en revenir au texte que nous examinons. Je voudrais d'abord rappeler que ce n'est pas la première fois qu'une telle PPL déposer sur le bureau des assemblées et parfois examiné en 2003 déjà, elle avait été adopté à l'Assemblée nationale mais jamais examiné au Sénat. La PPL que présente notre collègue il y a. Reprend dans le texte une même PPL déposée en 2018, on l'a dit tout à l'heure par notre collègue Éliane Assassi qui avait été examiné rejeté en séance le 20 novembre 2019. La rapporteure en était déjà notre collègue Muriel Jourda. Et je regrette qu'une concertation au sein de la commission des affaires sociales n'ait pas eu lieu avant le dépôt de cette PPL. D'autant qu'on peut légitimement s'interroger sur la nécessité de passer par un texte de loi. En effet la création de délégations touche à l'organisation interne des travaux de chaque assemblée. Ils n'ont pas il n'est pas nécessaire de légiférer sur de telles dispositions laissant les membres du bureau décidé dans la création ou non de cette délégation, c'est leur rôle. Il est vrai que la question des droits de l'enfant est un sujet transversal qui impacte de nombreux domaines tels que l'éducation, la santé, la justice la gouvernance. Vous le savez j'ai l'an passé était rapporteur de la loi du 8 février 2022 relatives à la protection des enfants. Nous avons constaté le manque d'efficience de cette politique au regard des moyens consacrés et avons fait des propositions concrètes. Certes, cette loi porte sur la protection des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. Mais au cours des nombreuses auditions que nous avons conduite tous les acteurs rencontrés particulièrement agissant auprès des enfants ont dit leur rattachement à la mise en place d'une veille pérenne et indépendante sur la question de l'élaboration de l'évaluation et du suivi des politiques publiques en faveur du droit des enfants. Je comprends qu'après la création au sein de l'Assemblée nationale d'une délégation aux droits des enfants. Ces associations demandent que le Sénat fasse de même. En effet, une délégation aux droits de l'enfant a été créée à l'Assemblée nationale le 13 septembre dernier sur décision de la conférence des présidents. Mais force est de constater que des sujets sur lesquels la délégation souhaite se pencher ont déjà largement été traité par le Sénat. Je ne le distrait pas tous ici, certains ont été conduits par la commission des affaires sociales. D'autre part, les commissions de la culture des lois de la commission des affaires économiques mais aussi par la délégation aux droits des femmes et je ne les rappellerai pas ici. Ainsi dans le profil de la révision constitutionnelle de 2008, c'est bien, via ses commissions permanentes que le Sénat exerce son pouvoir de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Il n'est peut être pas j'utile de multiplier les structures, le travail parlementaire ne s'en trouvera probablement pas plus efficace mais il convient que nos commissions particulièrement la commission des affaires sociales continuent de se saisir de ces questions, car de nouvelles formes de violence concomitante avec les usages de nos sociétés apparaissent. Madame la défenseure des droits et la CNIL ont récemment souligné l'urgence qu'il y a aujourd'hui à protéger les enfants des dangers du numérique. Je souhaite également que nous envisagions peut être via la création d'une mission d'information d'étudier la réalité de l'application des lois de 2007, de 2016 et de 2022 relatives à la protection de l'enfant qui ne sont pas également mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire et je sais Madame le Ministre ce que vous y êtes très attachés. Je sais, mes chers collègues qu'une société qui ne sait pas protéger ses enfants dans un monde apaisé rassurant est une société qui transige avec ses valeurs les plus fondamentales. Je vous remercie. Monsieur le président. Madame la secrétaire d'État madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues au sein de cet hémicycle, notre intérêt pour les droits de l'enfant est unanime. Notre volonté d'offrir à tous les enfants, les moyens de construire leur avenir demeure inaltérable et notre devoir d'éradiquer le fléau des violences qui leur sont faites. Quelles que soient les formes qu'elles peuvent revêtir est indéfectible. Pourtant en France et dans le monde les problématiques liées à l'enfance sont toujours d'une actualité brûlante. Et nombreux sont les défis qui restent à relever comme l'amélioration de la situation des enfants atteints de handicap ou du sort des enfants migrants aussi parce que la protection de l'enfant et son intérêt supérieur doivent être une préoccupation permanente du législateur. L'initiative de notre collègue Xavier Iacovelli mérite d'être salué. Et je félicite le groupe RDPI d'avoir inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour. Comme son titre l'indique, ce texte a pour objectif de constituer une délégation parlementaire aux droits de l'enfant. L'article unique institut en 1er lieu dans chaque assemblée. Une délégation parlementaire aux droits de l'enfant de 36 membres choisis à la représentation proportionnelle des groupes. En second lieu il charge ses délégations d'assurer le suivi de la politique des droits de l'enfant et leur permet d'être saisi de projets ou de propositions de loi, sur demande du Bureau d'une commission ou d'un président de groupe ou sur sa propre initiative. En 3ème lieu, il prévoit la remise d'un rapport d'activité annuel comprenant le cache échéant des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation. Enfin, il donne la possibilité à la délégation de l'Assemblée nationale et à celle du Sénat de décider de tenir des réunions communes une proposition de loi identique avait déjà été examiné au Sénat une première fois en 2019 et avait été repoussée. Or, depuis le 13 septembre dernier, l'Assemblée nationale s'est dotée d'une délégation aux droits des enfants. Composé de 36 membres. Cet élément nouveau nous incite à revoir notre position de 2019. En effet la création d'un équivalent au Sénat permettrait au cours de réunions menées conjointement de faire bénéficier la question des droits de l'enfant, de l'expertise des sénateurs, notamment à la lumière du rôle majeur que les collectivités territoriales jouent en faveur de l'enfance. Je pense notamment au département, chef de file des politiques sociales et de la protection de l'enfance.-- Par ailleurs, une délégation aux droits de l'enfant pourrait avoir un angle d'approche différent de celui des commissions permanentes qui effectue un remarquable travail logistique. Madame la secrétaire d'État. Chers collègues, la création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant faciliterait une démarche plus transversale pour traiter efficacement les multiples problématiques. Elle aurait aussi le mérite d'améliorer la connaissance des droits de l'enfant. Pas par les pouvoirs publics tout en donnant davantage de visibilité à ses droits. Pour toutes ces raisons, la majorité du groupe les indépendants votera en faveur de ce texte ce. Monsieur le président, madame la ministre madame le rapporteur, mes chers collègues. Nous le savons. L'enfer peut être pavée de bonnes intentions. Ainsi je crois utile de rappeler que la création d'une délégation relève d'usage du simple décision du bureau et je crois également utile de rappeler que la loi du 15 juin 2009. Ce n'est pas si vieux avait supprimé. Pas moins de 5 délégations dans un souci de rationalisation des travaux parlementaires.-- À vrai dire et c'est précis, en fait, cette proposition est surtout révélatrice. De ce que pourrait devenir notre vie parlementaire. Disons-le. Nous.-- Nous ne manquons pas d'outils pour nous emparer des enjeux de notre société. Il a bien sûr les propositions de loi et les amendements mais aussi les commissions d'enquête et les rapports d'information. Ainsi, plutôt que de se saisir de l'un d'eux aujourd'hui à cette heures nous discutons de la création d'une délégation plutôt que de débattre de solutions concrètes à des difficultés précise. J'ai bien conscience. Que cette proposition de loi peut se donner d'une certaine manière le bon rôle. Mais souvenez-vous, et j'en prends cet exemple quand j'en étais le co-rapporteur, que la commission des Lois et celle des affaires sociales à travers un rapport d'information conjoints ont pu pleinement s'investir sur le sort des mineurs dans. Par exemple et donc formulé de nombreuses propositions. Ce travail transversal sur des problématiques précises existent déjà et heureusement. En somme, je ne crois pas qu'imiter le travail parlementaire le rendra plus pertinent. Je ne suis d'ailleurs pas le seul puisque le groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat avait recommandé en 2015 18 et ne division trop importante de notre Champ de travail.-- En créant cette délégation. On se ferait plaisir. Je n'en doute pas, que l'on ne manquerait pas de communiquer dessus. Mais concrètement, rien ne changerait. Or, c'est le sens de mes propos. Le Parlement au vu des dernières abstention est attendu sur cette question, celle de la traduction de son travail dans le quotidien et français. Le travail parlementaire est reconnu pour sa qualité, c'est à mon sens indéniable mais les Français peut être comme l'auteur de cette proposition s'en lasse de voir nos rapports ne pas être pris en considération par un pouvoir exécutif qui pense. Seules les solutions n'a tous et connaître tout surtout. Admettons-le, c'est difficile à vivre. Lorsqu'on est dans l'opposition, mais je ne doute que le gouvernement puisse parfois entendre raison sur des dispositifs que nous l'encouragerions à mettre en place. Je milite donc pour un Sénat qui persiste à être véritablement une force de proposition. Plutôt qu'un Sénat qui se renfermerait sur lui-même et qui est, à l'instar de notre administration se perdrait dans une succession de comités Théodule et perdrait ainsi sa souplesse. Pour ces réseaux m'mes chers collègues. Je ne voterai pas cette proposition de loi. Ainsi qu'une grande majorité de mon groupe les républicains ce, ce vote n'est pas le le droit. Ce vote madame. La présidente. N'est pas contre les droits de l'enfant. Et je souhaiterais que certaines. Têtes hémicycle ne le réduise pas à une position caricaturale. Contre des enfants. En effet, nos travaux sénatoriaux démontre chaque jour le contraire. Je vous remercie.-- La discussion générale est Close. La commission n'a pas élaboré de projet de textile sont donc à la discussion de l'article unique de la proposition de loi dans sa forme initiale. Nous allons nous prononcer sur ce t'article qui vaudra en même temps vote sur l'ensemble de la proposition de loi et je vais maintenant solliciter les explications de vote. Donc que chacun se fasse connaître et chacune. J'ai vu d'abord Madame Guillotin.-- Merci monsieur le président. Alors en fait il existe, si j'ai bien suivi les débats une délégation aux droits de la femme une délégation aux entreprises, aux collectivités territoriales. Et bien d'autres et j'en passe. Donc c'est bien que le bureau du Sénat un moment a jugé, il a jugé qu'elle était utile et est capable de faire des choix. Cela est-ce que cela voudrait dire que les droits de l'enfant, eux ne mérite pas une délégation qu'il n'y a pas urgence à agir ou à s'emparer des des différentes problématiques. Je ne le crois pas puisque les différents travaux égrainés par la rapporteure nombreux ont montré qu'il avait un intérêt visiblement parce que le Sénat travaille sur ces sujets et l'excellent plaidoyer de monsieur Boon sur le le droit de l'enfant. En témoigne également alors si cette PPL. Peut permettre d'être le véhicule pour lever les freins visiblement. Que le bureau à faire de choix concernant les droits de l'enfant. Pour ma part en tout cas je pense je voterai pour évidemment cette PPL et j'incite. Tous ceux qui veulent s'emparer de sujets sociétaux au sein de cet hémicycle effectivement d'adopter et de voter pour cette PPL.

à chaque fois qu'il y a eu un débat ces derniers mois, ces dernières années dans notre pays, que ce soit sur le mariage pour tous sur l'adoption sur la PMA systématiquement les représentants de la majorité sénatoriale, ont mis en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Or aujourd'hui pendant que nous débattons de cette proposition de loi. Je voudrais d'abord regretter l'absence des collègues de la majorité sénatoriale qui ne sont pas présents alors que nous traitons justement des intérêts supérieurs de l'enfant. Première chose 2ème chose dans notre haute assemblée il y a les délégations, la délégation aux entrepris la délégation à la prospective. C'est faire injure à la commission des affaires économiques de laisser à penser qu'avant la création de cette délégation, personne ne travaillait ici sur les entreprises ni sur la prospective. Donc l'argument de Madame la rapporteure. Je ne le partage pas du tout, ce n'est pas parce que les commissions permanentes, travaille sur un sujet que cela interdit le Sénat, de créer une délégation spécifique. Enfin, je terminerai en disant que rendez-vous est pris pour dire que dans quelques mois ou dans quelques années, ce sera un membre ou une membre de la majorité sénatoriale qui proposera cette proposition de loi qui est la reprendra à son compte et à ce moment-là les conditions seront réunies pour réparer cette erreur que nous allons peut-être commettre aujourd'hui si nous votons majoritairement défavorablement à la commission à la proposition de notre collègue il y a Xavier Iacovelli que je veux remercier pour cette initiative. Suite, la parole est à madame Michèle Meunier. Si Monsieur le Président. Je voterai avec enthousiasme, cette proposition de loi en plus de tout ce qui vient d'être dit par nos collègues. Quand on dit souvent sur nos territoires à la fin d'une inauguration ou d'une rencontre concernant le secteur de l'enfance de la petite enfance quand on répète.-- Le proverbe africain. Il faut tout un village pour élever un enfant, soulignant par là et saluant le partenariat la coopération le travail ensemble le regard. Des différents acteurs qu'on retrouve sur le terrain de l'enfance. Je ne comprends pas et je trouve ça. Pas digne de notre haute assemblée de rater ce rendez-vous qu'on nous donne encore aujourd'hui avec le texte de Xavier Iacovelli. Donc je regrette et je déplore. et je déplore. Olivier Cadic pour une explication de vote.-- Si monsieur le président. Nouvellement élu au Sénat, je me souviens avoir interrogé en 2015. La secrétaire d'État en charge de la famille d'alors, notre collègue Laurence Rossignol. Le petit Bastien venait de mourir après avoir été mis dans le lave-linge par son père sur le mode essorage. Comme nous toutes et tous. J'avais été profondément bouleversé par ce drame, il mettait en lumière les carences d'un système qui avait failli à sauver un enfant d'une mort atroce. Je sais comme vous qu'il existe beaucoup d'autres Bastien et que nous peinons à recenser tous ces infanticides car il faudrait autopsié tous ces bébés morts prématurément de façon inexpliquée. La maltraitance des enfants ne s'arrête pas à nos frontières à l'étranger les familles françaises échappe parfois la protection de l'enfance. Certains enfants perdent parfois tout contact avec l'un de leurs parents comme nous l'avons souvent observé au Japon par exemple, grâce au travail de notre ancien collègue Richard Yung. Les consulats ne peuvent évidemment pas par faute de moyens et de formation. Être le prolongement de l'aide sociale à l'enfance, l'aide aux victimes de violences notamment familial et néanmoins développé petit à petit c'est à notre capacité à protéger les plus faibles qu'on reconnaît une société civilisée. Avant de pouvoir agir, il faut connaître et mesurer l'ampleur du problème. Le système mis en place pour y faire face. La création d'une délégation aux droits de l'enfant qui consacrera ses travaux à améliorer la protection des enfants me semble impérieuse. Je salue cette initiative de notre collègue Xavier il Iacovelli. Je le remercie d'avoir cité d'ailleurs la proposition précédente de la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam qui comme moi représente les Français établis hors de France Avec le même enthousiasme que certains collègues. Cette proposition de loi, je vous remercie. Monsieur le président, madame Nice madame la rapporteure, chers collègues.-- Je remercie déjà tous ceux qui ont pris la parole pour soutenir cette proposition de loi je reprends également les mots de du sénateur Burgy sénateur Cadic. Sénatrice Meunier, merci pour pour ses mots et je je souscris complètement à, à, aux propos que vous avez tenus. je voudrais juste reprendre quelques mots sur sur le mépris, pardonnez-moi, dans ce moment un peu sympa. Le mépris qui ont été affichés sur l'affichage sur une proposition du coeur. Non en fait je pense que au contraire c'est une proposition de raison. C'est une proposition de raisons et notamment en nous appuyant sur l'argumentaire de la qui a listé un certain nombre de travaux d'audition et et de. Et et de rapports Odysseum rapport qui ne font pas forcément une loi hein. Je vous rappelle mais audition et rappeur qui justement montrent que nos travaux sont. Sont nombreux au Sénat et que nous avons besoin de coordonner et d'avoir quelque chose de transversal, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans le mépris et donner dénaturer les travaux des parlementaires et des initiatives parlementaires pour afficher peut être quelque chose sur lequel vous êtes peut-être mal à l'aise sur votre position. Je peux le comprendre mais en l'occurrence. C'est c'est ce je pense qu'on peut on n'est pas obligé d'aller dans le mépris. Après je j'en compte j'entendais aussi la question de la temporalité, alors je l'ai entendu dans cet hémicycle. Je l'ai entendu aussi dans les couloirs de cet hémicycle sur la tempe, l'arrêter, vous vous rendez compte, on va pas créer une délégation à 9 mois des renouvellement sénatorial et imaginez-vous qu'on pourrait s'en servir. Parce que c'est quand même porté par l'opposition sénatoriale sincèrement engageons-nous ici. Si le problème il est de, de faire cette délégation en septembre ou en octobre 2023. Engageons nous ici il y a pas de souci moi tant que la délégation. Et créé on peut attendre 2023 pour la créer. Mais nous n'arrêtons pas sur une question de temporalité. On est sur le droit des enfants, on n'est pas sur une question électorale et partisane Moi, je reprends les arguments du sénateur bonne qui qui malheureusement est est parti il disait oui je pense qu'il faut le faire dans le cadre de la commission des affaires sociales peut être créé un groupe d'étude dans le cadre. Oui ben très bien, c'est ce que j'ai demandé en 2020. Ça m'a été refusé, enfin je veux bien qu'on ait le débat mais on peut avoir le débat régulièrement si à chaque fois on refuse quand on fait des propositions. Ne vous étonnez pas qu'on passe dans l'hémicycle, au bout d'un moment pour demander l'avis des parlementaires. J'espère juste en tout cas que les consignes de vote seront respectées. Parce que moi j'ai eu beaucoup de soutien de tous les groupes y compris de la majorité sénatoriale que je vous remercie. Je prends comprend que on étant j'ai dit c'est difficile pour certains d'être présents. Dans l'hémicycle que beaucoup soutiennent cette proposition de loi et en tout cas j'invite tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ont les délégations de vote de voter correctement pour pour cette proposition de loi et de voter favorablement. Merci. Madame la rapporteure et les représentants de la majorité à l'LR sénatoriale nous ont invités à parler non pas des droits de l'enfant mais de fonctionnement du Sénat. Alors c'est du fonctionnement du Sénat. Je vais dont je vais vous parler dans ma mon explication de vote. Je me suis suffisamment exprimé sur la délégation.

ils sont hostiles. Sur les 8 groupes du Sénat six sont favorables à cette proposition de loi. Un groupe est partagé et un groupe il est majoritairement hostile et par notre système de vote.-- Par vote par scrutin public malgré les chiffres que je viens de donner. Il est possible que dans quelques instants cette proposition de loi soit rejeté. Alors si vous voulez parler du fonctionnement du Sénat. Je vous suggère là un beau sujet c'est le respect du vote dans le Sénat.

Et donc Madame Dindar souhaite encore ajouté une explication de vote. Mais. Merci monsieur le président, je suis désolé, j'avais demandé la parole, j'avais levé la main, moi je suis très favorable et je voterai pour cette proposition de loi. D'abord parce que je crois que les départements eux-mêmes. attendent que nous travaillons sur ce sujet et puis. À la Réunion, l'université vient d'organiser avec. Le conseil départemental avec l'ensemble des associations. De la zone de l'océan Indien. Il y avait là aussi des représentants de Mayotte, un grand colloque sur les droits des enfants pour. Donner des chiffres qui sont très alarmants principalement sur la scolarité des enfants sur la méconnaissance des mamans sur les grossesses précoces. Alors, vous comprenez. Oui, vous comprendrez que que moi je suis personnellement favorable mais je dirai à mon. Nami Xavier que il n'y a pas de mépris pour en avoir discuté avec bon nombre de mes collègues de la part du groupe centriste. Beaucoup mettent surtout la forme plus qu'au niveau du fond et donc. C'est peut-être pour cela que certains s'abstiendront ou voteront contre. Et donc je voulais quand même faire écho de toute la discussion que j'avais eu personnellement avec beaucoup de mes collègues.-- Monsieur le Président Madame le Ministre. Je remercie Madame Dindar puisque le propos pouvaient tenir était à peu près celui que je voulais tenir. Car lorsque l'on parle de mépris. De la majorité sénatoriale puisque disons les choses, c'est c'est ce que vous avez dit. On ne peut pas l'entendre. Pas plus qu'on ne peut entendre que le fond, la forme cacherait le fond parce que nous aurions un désintérêt pour la protection des enfants, je n'étais pas là en début de séance, je m'en excuse. Il a été dit, ici dans cet hémicycle, que la forme cachait le fond. Et, laissant entendre par ailleurs que les gens. De la majorité sénatoriale. En réalité ce fichet je fais très court, de l'intérêt des enfants. Je vous rappelle quand même que il a été rappelé le nombre de travaux qui ont été fait le dernier d'entre eux d'ailleurs et celui sur les agressions sexuelles des mineurs. Ils nous ont fait un très gros travail à la commission des lois et on a amélioré la défense évidemment heureusement des enfants. La question ne se pose pas sur le fond elle se pose sur la fin, je ne suis pas défensif. Je n'ai je n'aime pas Madame. La Ministre Rossignol. Les procès d'intention. Je n'aime pas les procès d'intention. C'est déjà le cas. À plusieurs à plusieurs. Dans plusieurs débats. Je n'aime pas les procès d'intention on peut divergent, certains sujets mais les procès d'intention sont pour moi pas acceptable, c'est simplement ce que je vais vous dire,

L'avis de la commission étant donc défavorable et l'avis du gouvernement étant un avis de sagesse. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56, le scrutin est ouvert.

Ça ne demande plus à voter. Le scrutin est clos. Résultat. Votants 345. Exprimés. 331. Pour 153. Contre 178. Le Sénat n'a pas adopté. C'est pour ça que la l'annonce faisant foi et celle que je viens de prononcer que je répète. Que je répète votants 345. Exprimés 331. Pour 153. Contre 178, le Sénat n'a donc pas adopter. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise. À 16h, pour l'examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée. Visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves. La séance est suspendue.